l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français, présenté par Madame Josiane Costes et plusieurs de ses collègues notre séance se déroule dans des conditions de respect des règles sanitaires mises en. En place depuis le mois de mars, l'hémicycle, fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant et après chaque séance, les micros seront désinfecté après chaque intervention, j'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité, je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'est effectuée par les portes situées au pourtour de l'hémicycle, je rappelle que tous les orateurs, y compris le gouvernement s'exprimeront depuis leur place sont montés à la tribune je rappelle enfin qu'afin de limiter la circulation de documents, vous êtes invités à utiliser vos tablettes et la fonctionnaire l'IT en séance sur notre site Internet pour prendre connaissance du des rouleurs et des amendements, des liasses resteront à votre disposition, à la demande dans la discussion générale, la parole est à Madame Josiane Costes, auteur de la proposition de loi et vous avez 10 minutes chers collègues. Merci madame la présidente. Madame, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me réjouis que nous puissions discuter aujourd'hui de ce sujet vital, et qu'il n'ait pas été remis à plus tard, du fait de la crise sanitaire qui a touché notre pays, au contraire, comme l'ont souligné, beaucoup d'observateurs, et notamment le défenseur des droits : le confinement a rendu les inégalités familial plus perceptible le déconfinement représente également un nouvel enjeu pour les services sociaux, après 2 mois de Liens distendus avec les mineurs placés à l'issue de mon expérience de professeur et à la suite des auditions et des visites que j'ai eu l'occasion de mener en tant que sénatrice cette proposition de loi s'adresse à 2 types de vie de vulnérabilité chez l'enfant,

les tranches d'âge, de toutes les tranches d'âge, la seconde est plus récente et elle résulte de l'isolement d'adolescents envoyés en France à la suite d'un projet familial construit autour et pour eux, ces 2 cas de figure, ont en commun de bouleverser le développement de l'enfant en le mettant face à des choix et des responsabilités inadapté à la maturité communément admise à son âge, ces 2 types de vulnérabilité présente également des défis inégaux dans mon département, dont nous connaissons les limites budgétaires. Inévitablement, les déséquilibres démographiques sur notre territoire se traduisent également par des dépenses très variable d'un dans le département à l'autre à l'échelle nationale, les besoins de la protection de l'enfance d'ont cessé de croître ces dernières décennies, à la fois parce que nos exigences de protection ont augmenté, ce qui est positif, mais également avec l'émergence de nouveaux profils de mineurs vulnérables tels les mineurs isolés étrangers que j'évoquais, ils seraient près de 40000 aujourd'hui pour 300000 enfants concernés par l'ASE, il me paraît nécessaire que nos institutions s'adapte à cette réalité sociale que nous ne pouvons continuer à ignorer en formulant ses propositions, nous nous sommes donc attachés à nous départir de tout dogmatisme à ne pas juger les circonstances qui ont produit ces vulnérabilités mais simplement à constater leur existence et à tenter de concevoir les outils pragmatique destiné à pallier chacune d'entre elles, l'histoire est une galerie de tableaux il y a peu d'originaux et beaucoup de copies, écrivait Tocqueville, beaucoup de ces propositions reprennent des pistes déjà évoquées dans le passé, en les approfondissant, il y a, on les a en les associant pour former une stratégie cohérente autour du renforcement du du recours à l'adoption simple qui est au coeur du dispositif à l'article 3 jusqu'à présent, la politique française de l'aide sociale à l'enfance s'articule autour d'une attaque d'une alternative qui ne pas qui ne me paraît pas satisfaisante soit la préservation des Liens biologiques exclusif soit l'adoption plénière et l'effacement de ses Liens biologiques cette dichotomie forte me semble de nature à accroître le dilemme de des adultes accompagnant l'enfant juge assistant social, conseil de famille pour une raison qui m'échappe, l'adoption simple continue d'être une forme très peu, alors qu'elle existe depuis 1804 la loi de 2016 la récemment réformé pour prévoir qu'elle ne peut être révoquée qu'à la majorité de l'individu, contrairement à l'adoption plénière le lien avec la famille biologique est donc maintenu l'adopter peut en conserver le nom auquel s'ajoute celui de la famille adoptante la famille biologique d'origine conserve d'ailleurs l'obligation de le nourrir, dans le cas où la famille adoptante ne pourrait plus y subvenir pour le parent biologique, pardon, cette solution pourrait s'avérer moins déchirantes et permettre une meilleure coopération avec les services sociaux l'adoption simple permet, qui plus est d'établir des Liens juridiques plus durable et plus étoffés qu'entre le mineur est une famille d'accueil rétribués pour cela ou un tiers digne de confiance dont l'enfant ne porte pas le patronyme et qui ne se double pas nécessairement d'une délégation de l'autorité parentale, la superposition des Liens biologiques et de nouveaux Liens Zappa affectif me paraît être là me paraît être la plus ça même de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, enfin parce qu'elle repose sur la gratuité, elle s'avère également relativement économique les articles 1 à 4 s'inscrivent dans la logique de recherche d'une plus grande stabilité pour l'enfant, cette même logique qui avait prévalu en 2016 avec la redéfinition du projet de l'enfant et l'inscription de la recherche de stabilité au sein des missions de l'ASE, il s'agit en particulier d'adapter les procédures à l'âge de l'enfant en fonction du risque d'impact pour son développement et de lui apporter le plus rapidement possible une solution stable qui ne soit pas totalement excluante pour la famille biologique madame et monsieur les rapporteurs, je comprends la prudence, faute de données suffisantes sur les évolutions de la loi de 2016, j'espérais justement que cette initiative permettrait d'en obtenir davantage dans cette proposition de loi les mineurs isolés étrangers prennent une place particulière, comme je l'évoquais plus tôt au regard des données disponibles, leur situation semble différente des autres mineurs concernés par l'ASE, il est vrai que pour ces adolescents leur parcours migratoire peut les amener à une maturité plus précoce que des enfants élevés dans des quatre protecteur, ce qui justifie pour certains de ne pas les prendre en charge d'une certaine manière, leur situation se rapproche de celle de jeunes majeurs issus de l'ASE que notre proposition de loi propose également de mieux accompagner, nous savons qu'en réalité la majorité est une fiction législatives qui est d'ailleurs passée de 21 à 18 ans en 1974 par la seule volonté du législateur ainsi au regard de notre droit, nous ne pouvons nous dispenser de les considérer encore comme des enfants de leur offrir la protection que la minorité garantie, sauf à introduire des ruptures d'inégalité basé sur le seul critère de nationalité, ce qui n'est pas acceptable, nous savons aujourd'hui que notre inaction les expose à des réseaux à de la violence et leur errance nourrit un climat d'insécurité qui ne convient à aucun d'entre nous, en particulier leur difficulté d'ouvrir un compte bancaire renforcent leur vulnérabilité en les contraignant de conserver leur argent en liquide avec eux, l'un d'entre eux est mort en février, en tentant de conserver son pécule, tous ceux qui ont accompagné ces jeunes savent à quel point la reconnaissance est un vecteur 20 vertueux d'intégration, c'est pourquoi je propose quelques simplifications administratives destinées à leur permettre de s'insérer plus facilement dans notre société je ne néglige pas l'importance de l'effort budgétaire que ces mesures représentent pour nos concitoyens, mais je pense que la société Sanchis s'enrichir et de la sensibilité de ses enfants et de ces jeunes au au parcours moins rectiligne que bon nombres d'entre nous et que nous avons beaucoup à apprendre de leur résilience, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur à la rapporteur de la commission des lois, et vous avez 10 minutes chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, les sujets abordés par la proposition de loi que nous examinons sont tous d'actualité, notre collègue Josiane Costes participe ainsi à une large réflexion menée sur la politique publique en matière de protection de l'enfance, dont chacun s'accorde à dire qu'elle doit être améliorée, de nombreux travaux ont été publiés au cours des derniers mois, je citerai parmi eux, le rapport sur l'adoption de notre collègue Corinne Imbert et de la députée Monique Limon remis en octobre 2019, ou encore à l'avis du comité consultatif national d'éthique, publié le 7 mai de son côté, le gouvernement et vous, monsieur le ministre avait lancé une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour les années 2019, 2022 qui est principalement fondée sur une contractualisation pluriannuelle entre l'État et les départements, elle comprend aussi un volet qui devrait être mis en oeuvre par voie législative, en particulier sur l'adoption. Monsieur le Ministre, peut-être pourrez-vous nous faire un point de son calendrier. Par ailleurs, la crise du Covid 19 et le confinement qui ça n'est suivi ont mis en lumière avec acuité la difficile situation des enfants victimes de violences intrafamiliales et de ceux qui vivent dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance ou dans des familles d'accueil, la proposition de loi se fonde sur un certain nombre de constats et d'objectifs partagés par les auteurs des travaux précédemment évoquées et comprend de nombreuses mesures toutefois, il nous a semblé que le texte initial n'apportait pas de réponse suffisamment efficace et globale aux problèmes actuels, c'est pourquoi la commission des lois n'a pas adopté de texte, je vais vous présenter brièvement ses articles, étant précisé que les articles 5 6 et 9 ont été délégués au fond à la commission des affaires sociales, les articles 1 et 2 visait à accélérer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental dans le but d'offrir le plus tôt possible une prise en charge pérenne des enfants via l'adoption, l'article 1, permettrait de constater le délaissement au bout de 6 mois seulement et non plus un an pour les enfants âgés de moins de 3 ans, l'article 2 supprimerait l'obligation préalable de proposer des mesures de soutien appropriés aux parents, il imposerait également aux tribunaux judiciaires de statuer dans un délai de 2 mois, réduite moi si l'à moins de 3 ans à compter du dépôt de la requête, la commission des lois jugées trop hâtif le postulat selon lequel accélérer la procédure de délaissement parental améliorerait automatiquement l'adaptabilité des enfants tous les enfants délaissés ne devienne pas pupilles de l'État et toutes les pupilles de l'État ne sont pas nécessairement adoptables par ailleurs, le délai d'un an pour constater le délaissement semble raisonnable au regard des difficultés que traverse des familles concernées, le fait de devoir proposer aux parents des mesures de soutien approprié pendant cette période et respectueux de l'article du 18 de la convention internationale des droits de l'enfant et permet de mieux caractériser ensuite l'absence d'implication des parents à contraindre les juges à statuer dans un délai de 2 ou un mois ne semble ni réaliste ni souhaitable au vu de la complexité et des enjeux de ce dossier et de la nécessité de procéder à des investigations sur l'article 3 qui concerne le procès-verbal de remise de lymphome par ses parents au service de l'ASE notre collègue Josiane Costes propose une nouvelle rédaction qui nous a semblé pouvoir être adopté, nous l'examinerons tout à l'heure, l'article 4 tend à rendre plus difficile de la reprise de l'enfant, placés à l'initiative de l'un ou de ses parents auprès des services de l'âge pendant la période de réflexion de 2 mois, qui leur est accordé 2 formalités seraient imposé un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille dont il n'est pas précisé s'il aurait la possibilité de s'opposer à la restitution de leur enfant, ce dispositif nous a paru susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale, la durée de réflexion est déjà suffisamment brève, sans qu'il soit besoin sans doute d'y ajouter des obstacles, l'article 7 vise à étendre dans tous les départements, la validité de l'agrément délivré pour l'adoption des pupilles de l'État par un président de conseil départemental, il est à craindre que la multiplication des candidatures enregistrées auprès des conseils départementaux aboutissent à une surcharge administrative pour leurs services, il vaudrait mieux faciliter les échanges au niveau national entre conseils départementaux, en particulier lorsqu'il s'agit d'un fan dits à besoins spécifiques, c'est-à-dire porteurs de pathologies ou de handicap plus âgés ou encore Membre de fratrie qui représentent près de la moitié des pupilles de l'État mais correspondent rarement aux attentes des parents candidats à l'adoption, notre collègue Josiane Costes propose d'ailleurs à ce sujet un amendement permettant d'asseoir juridiquement un fichier national désagrément qui nous semble intéressant l'article 8 vise à créer un mécanisme de coordination en matière de parrainage d'enfants étrangers, mais la commission des lois relever diverses difficultés dont une absence de définition légale du parrainage international, l'article 10 vise à instaurer une présomption de désintérêt à l'égard des parents de mineurs étrangers arrivés sur le territoire national et qui se trouveraient isolé pour faciliter la délégation de leur autorité parentale, outre le fait que les textes en vigueur permettent déjà aux juges de prononcer le délégation d'autorité parentale pour un mineur isolé étranger quand c'est nécessaire, je dis : ce dispositif pardon nous est apparu attentatoire au droit des parents de ces enfants qui souvent suivent de près le parcours migratoire de leur enfant et ne sont donc pas tous, délaissant l'article 11 attentats à permettre l'attribution automatique de nationalité française aux mineurs adoptée informe simple et donc dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues pour l'adoption plénière cette nouvelle modalités d'octroi de la nationalité ne semble pas nécessaire pour faciliter l'intégration de ces mineurs qui dispose d'une voie spéciale a d'accès à la nationalité, de plus, une telle mesure opérerait un renversement très importante dans notre droit et modifierait la nature même de l'adoption simple l'article 12 vise à transférer au juge des enfants, la compétence pour statuer sur une mesure de délégation d'autorité parentale à un tiers concernant les mineurs isolés étrangers toutefois le juge aux affaires familiales et le juge naturel de l'autorité parentale et la commission des lois n'a pas trouvé opportun de prévoir une dérogation qui serait limité à un seul groupe d'enfants, les mineurs isolés et dans le cadre d'une seule procédure celle relative à l'autorité parentale, l'article 13 concernent le droit au compte en banque à tout mineurs étrangers dont les parents ne réside pas sur le sol français, l'auteur de la proposition de loi propose une nouvelle rédaction de et la Commission s'y est déclaré favorable, nous le verrons tout à l'heure, l'article 14 vise à prévoir à la délivrance obligatoire d'un certificat d'authentification de titres d'identité par les services des douanes lors d'un 1er contrôle pour simplifier, démarches administratives, des mineurs isolés étrangers c'est très innovant, mais ça ne semble ni opération éléments possible, ni juridiquement souhaitables en tout état de cause, je le droit existant prévoit déjà qu'en cas de doute sur l'état civil de mineurs non accompagnés, confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est au préfet qu'il appartienne renverser par tout moyen la présomption de validité qui bénéficie aux actes d'état civil étranger, l'article 15 tendent à faciliter l'admission exceptionnelle au séjour des mineurs isolés qui ont été recueillis par l'ASE après leur 16 ans et intégré dans des cursus professionnalisant, il ne nous semble pourtant pas opportun de supprimer le caractère exceptionnel de la délivrance de ce type de titres ni de dispenser ces mineurs de la condition de suivre une formation de 6 mois au moins l'admission exceptionnelle au séjour doit rester une compétence discrétionnaire du préfet limitée et appréciée au cas par cas en fonction des perspectives concrètes d'intégration des enfants étrangers concernés. La commission des lois vous invite donc adopter les articles 3 et 13 au bénéfice des amendements proposés par notre collègue Josiane Costes qui a utilement retravailler la rédaction, nous pourrons également adopté 2 articles additionnels, en revanche, la commission des lois vous proposera de supprimer ou de ne pas adopter les autres articles de cette proposition de loi, à titre personnel, je souhaiterais dire et qu'il y a un point qui me semble particulièrement bloquant pour réformer le droit existant, c'est notre manque de recul sur les différents dispositifs en place et leurs effets à long terme, d'ailleurs, Madame Coste l'a dit tout à l'heure et le même dans ses propos, il n'y a pas assez de connaissances, de travaux de recherche menée dans la durée, sur des cohortes d'enfants ce qu'on appelle des études longitudinales, il est très difficile de connaître de manière statistique et qualitative, les parcours en protection de l'enfance des enfants afin de comprendre quelle peut être la conséquence de telle ou telle décision les concernant, notamment en termes de délinquance de scolarité, nous ne connaissons malheureusement que les cas dans lesquels les choses se sont très mal passées, je rappellerai pour conclure les propos de la présidente du groupement d'intérêt public Enfance en danger, qui me semble très vrai l'indignation et les émotions suscitées par toutes les situations difficiles vécues par les enfants de la protection de l'enfance se constituent des moteurs puissants de l'action, mais il est malgré tout nécessaire de leur adjoindre connaissance et méthode. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Josiane Costes, dont je salue le travail et l'engagement sans faille sur le sujet des mineurs vulnérables nous permet de discuter aujourd'hui de la protection de l'enfance qui doit retenir toute notre attention, en particulier dans le contexte actuel de pandémie que nous traversons. La commission des affaires sociales à examiner au fond les articles 5 6 et 9 qui concerne l'aide sociale à l'enfance, les services de l'aide sociale à l'enfance sont de plus en plus sollicités, le nombre de mesures de suivi ayant augmenté de plus de 30 % en 20 ans, soit 344000 mesures d'azote étaient ainsi en cours auprès des mineurs et jeunes majeurs en 2017, dont la moitié pour un placement la crise sanitaire rappelle en outre la nécessité de mieux protéger les enfants en particulier contre les violences intrafamiliales auxquels ils sont davantage exposées depuis le confinement cette situation nous impose de renforcer la prévention et la prise en charge des mineurs vulnérables dont ceux victimes de maltraitance ou de carences éducatives, il existe malheureusement une certaine hétérogénéité dans l'accompagnement des mineurs et jeunes majeurs par l'ASE selon les départements, bien souvent par manque de moyens, c'est ce que j'ai pu constater pour l'examen de l'article 6 de cette proposition de loi cet article propose de rendre obligatoire la prise en charge par l'ASE de mineurs émancipés et 2 majeurs de moins de 21 ans, en situation de vulnérabilité. Cet accompagnement qui prend aujourd'hui la forme d'un contrat jeune majeur est à l'appréciation des conseils départementaux, la commission a émis plusieurs réserves sur la mesure proposée qui risque d'une part, de créer d'importantes dépenses non compensées pour les départements, au risque de diluer les moyens consacrés à la d'autre part, il apparaît préférable de conserver une forme de souplesse pour l'accompagnement des jeunes majeurs selon les besoins de chacun, tous les jeunes majeurs, suivie par la zone n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement jusqu'à 21 ans, et non pas forcément le souhait d'être accompagné jusque 21 ans, un travail sur la lutte contre les sorties sèches par contre de l'ASE comme s'y emploie le gouvernement en lien avec les départements, nous paraît préférable à l'instauration d'une obligation quant à l'article 9, il propose que les allocations familiales dues au titre d'un enfant, confie à l'ASE ne puissent être maintenus que partiellement à la famille, sur décision du juge, je rappelle que le principe posé par la loi et celui du versement au service de l'ASE des allocations familiales dues au titre d'un enfant placé par dérogation, la loi prévoit toutefois que pour les situations de placement judiciaire, le juge peut décider de maintenir ses allocations à la famille si celle-ci participent à la prise en charge morale ou la prise en charge matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter son retour dans le foyer, le maintien des allocations à la famille et donc laissée à l'appréciation du juge, en pratique, il ressort des quelques chiffres obtenus qu'il n'est pas systématiquement déroger au principe du versement à l'ASE, des chiffres qui avaient été communiquées par le gouvernement en 2016 faisait état d'un versement à l'ASE pour 45 % des situations et d'un maintien des allocations familiales à la famille pour 55 % des cas j'ajoute que dans certaines situations, il ne paraît pas opportun que ces allocations soient retirés à la famille par exemple, dans les cas de placement en urgence de courte durée, les placements au titre de l'enfance délinquante ou encore pour les familles nombreuses ou des Liens sont encore maintenus avec l'enfant, pour ces raisons, la commission a considéré qu'il était préférable de laisser au juge une certaine marge d'appréciation pour s'adapter aux différentes situations familiales au total, il me semble que certains n'équilibre soit opérée entre maintien et retrait des prestations aux familles ayant un enfant placé, je rappelle à ce propos que depuis la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, l'allocation de rentrée scolaire n'est plus versée à la famille de l'enfant, confiés à l'ASE elle est reversé à cette enfance sous la forme d'un pécule lorsqu'il atteint sa majorité pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires sociales n'a pas adopté les articles 5 6 et 9 de la proposition de loi nous en nous entamons donc notre discussion sur la base du texte initial déposé par notre collègue Josiane Costes, l'examen de ce texte est aussi l'occasion d'échanger sur les voies d'amélioration de la protection de l'enfance qui connaît encore de trop nombreuses insuffisances le ministre pourra certainement nous préciser les mesures en cours de déploiement en faveur des mineurs en danger dans le cadre de la stratégie pour la protection de l'enfance, mise en place par le gouvernement à l'Automne dernier, vous pouvez aussi Monsieur le Ministre, nous indiquer quelles mesures sont engagées ou envisagées, pour soutenir les acteurs de la protection de l'enfance, en particulier les familles d'accueil dans le contexte de la crise sanitaire, nous devons leur apporter sans tarder les moyens de poursuivent leur mission pour protéger et accompagner les mineurs vulnérables, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités, de la santé. Merci madame la présidente. Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure. Madame la sénatrice. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Il y a toujours de notre enfance, un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir. Ces mots de l'écrivain britannique Graham Greene, me semble être en parfaite résonance avec l'objet de la proposition de loi. Donc, nous allons discuter ce jour, c'est au moins l'occasion je vous en remercie pour cela de mettre dans la lumière, ces enfants, ces jeunes pour lesquels les portes restent trop souvent fermé. Je sais, Madame la sénatrice, que ces sujets vous tiennent particulièrement à coeur, c'est un sujet qui fera forcément écho dans votre assemblée, non seulement parce qu'il siège de nombreux ancien président ou présidente vice-présidents ou vice-présidents de conseils départementaux qui ont oeuvré sur leur territoire pour protéger au mieux les enfants, les jeunes les plus vulnérables, mais aussi parce que votre hémicycle compte d'anciens ministres qui ont été en charge de dossiers relatifs à l'enfance comme le président. Qui a porté la loi du 5 mars et la ministre Rossignol qui, s'appuyant sur le travail remarquable des sénatrices Meunier et Dini a défendu la loi du 14 mars 2016. Je peux enfin citer les initiatives et travaux menés. Par la sénatrice Imbert, j'y reviendrai évidemment et par le sénateur Yachvili plus récemment au printemps 2019 nous avons tous évidemment collectivement un devoir de protection vis-à-vis de ces jeunes dans la trajectoire de vie est plus difficile et parfois dramatique, c'est la mission de notre service public de d'aide sociale en France avec près de 340000 enfants et jeunes accompagnés dans des lieux d'accueil au domicile familial, et que ce soit ici l'occasion aujourd'hui pour moi de saluer saluer une nouvelle fois publiquement l'engagement des élus départementaux de l'ensemble de leur équipe mais aussi des travailleurs sociaux, des assistants familiaux, des associations, des établissements et des services. Ces derniers sont quotidiennement auprès de nos enfants et ils l'ont été plus encore au cours de cette crise. Mais, au-delà, d'assurer leur protection et leur sécurité, nous devons aussi les accompagner vers l'autonomie. Et c'est d'ailleurs ce à quoi fait explicitement référence votre proposition de loi, Madame la sénatrice, quand vous parlez d'épanouissement et de développement. Dans son titre, et quand on connaît les chiffres effectivement certaines études. Certaines enquêtes, quand on sait par exemple que dans certains territoires 40 % des enfants placés ont un parent qui lui-même a été placé. Quand on sait que 25 % des jeunes. Sans domicile fixe ont eu à un moment de leur vie, un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Que 20 % des adultes qui sont en détention ont aussi connu un moment l'aide sociale à l'enfance. On se rend bien compte que nous sommes encore loin d'avoir brisé ce qui semble s'apparenter à une chaîne de fatalité. Ses enfants et ses jeunes protégés ne demande qu'à être des enfants comme les autres en réalité. être considéré aussi comme des enfants comme les autres, rien de plus, rien de moins, j'en suis convaincu. Et c'est tout ce qu'ils nous demandent c'est tout ce que nous leur devons mais c'est tout le sens de l'action que je mène depuis 16 mois. Et je vais effectivement prendre cette occasion pour vous préciser quelques-uns des quelques-unes des des mesures qui ont été engagées dès ma nomination, c'est l'a été rappelé par. Les rapporteurs j'initient une large concertation avec l'Assemblée des départements de France, l'ensemble des acteurs associatifs et institutionnels 6 groupes de travail où avait été installé pour aboutir, 4 mois après à une stratégie de prévention et de protection de l'enfance, et ce n'est pas totalement innocent évidemment d'avoir intégré la notion de prévention dans le titre est au coeur de cette stratégie, pour les 3 prochaines années, alors oui, cette stratégie porte, d'une part, l'ambition d'un partenariat renouvelé entre l'État, les collectivités départementales qui sont chef de file. La protection de l'enfance, depuis les lois de décentralisation, et c'est pour ça que j'ai défendu à l'instar de ce qui avait été initiée pour la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, définie par le président de la République et le gouvernement en septembre 2018 d'une contractualisation sur la base d'engagements communs réciproque. Et c'est autour de 4 objectifs d'une part, agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille, donc c'est tout ce volet prévention insuffisante dans notre pays, quel que soit le Champ et dans le Champ social, en particulier sécurisé ensuite les parcours des enfants protéger et prévenir les ruptures oui ce sont des enfants qui connaissent des ruptures de vie. Et dont le système va lui-même généré de multiples ruptures. Pouvant s'apparenter à une forme de maltraitance institutionnelle dans certains cas, ça ce n'est pas admissible et nous devons faire en sorte de sécuriser ces parcours d'éviter ces ruptures : donner aux enfants les moyens d'agir et de garantir leurs droits. La pleine participation des enfants à l'élaboration de cette politique publique dans nos instances de gouvernance, j'y reviendrai, doit être un objectif, tout comme la pleine participation des enfants à leurs conditions de vie. à la façon dont ça se passe concrètement dans leurs établissements dans leur famille, dans les conseils de vie sociale doit aussi être renforcée. Enfin, préparer leur avenir sécuriser leur vie d'adulte. En articulation je reviendrai là aussi avec les mesures de stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui dès dès avant ma nomination. Prévoyait déjà. De s'attaquer à la question des sorties dites sèches. Cette démarche les proposer à l'ensemble des départements. En un mois, plus de 60 départements ont répondu favorablement. Avec des propositions très concrètes des projets très élaboré, tant sur le volet prévention, je pense notamment à la PMI qui faisait partie d'ailleurs des obligations en quelque sorte, vous m'excuserez du terme vous savez proposé au département, ce que nous avons besoin de renforcer ce toutes formidable outil qu'est la PMI, mais aussi pour ce qui est protection de l'enfance, et je pense notamment à tout le volet de l'accompagnement médico- social des enfants de l'aide sociale à l'enfance, vous le savez. Plus de 20 % des enfants de l'aide sociale en France ont une reconnaissance MDPH sont en situation de handicap et l'articulation de dispositifs sociaux et médico-sociaux. Dans notre pays, qui aime bien encore fonctionner en silos. quand vous êtes un usager qui est au croisement de politiques publiques et de disques de dispositifs dans notre pays, trop souvent encore, manque de pot, vous tombez dans le trou qui est entre les 2. Et d'ailleurs, période de confinement et de crise dont nous sortons progressivement a mis à l'épreuve. Cette articulation. Ou ses défauts d'articulation. à imposer aux acteurs d'être particulièrement créatif pour assurer une continuité de prise en charge dans cette période qui était compliqué pour tout le monde, chacun, de toute façon, a dû faire montre d'adaptation et de créativité, mais il y a beaucoup mieux et plus à faire et c'est au coeur de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance que je porte et ça a été au coeur des projets que nous ont remonté les départements 30 d'entre eux vont l'initier dès cette année. La semaine dernière, nous avons signé et publié, avec Olivier Véran la circulaire qui fixe le cadre opérationnel des discussions à l'attention des préfets, des directeurs généraux des ARS et des départements et qui va donc permettre dans les prochains jours, semaine, enfin en tout cas, Rennes ne s'y oppose plus. à ce que soient délégués de façon très concrète les 80 millions d'euros que vous aviez voté dans le cadre du Plfss et du PLF 2 l'année dernière. Au-delà de ces 30 départements. Viendront. L'intégralité je l'espère, des départements, par la suite, puisque notre stratégie, a évidemment vocation à s'étendre à tous. Malgré la crise sanitaire que nous traversons encore et face à laquelle les départements ont été et reste en première ligne cette contractualisation et donc d'ores et déjà relancé, et il le fallait, il y avait urgence à agir alors contrairement à ce que certains feignent de croire essaye de laisser croire cette stratégie nationale ne se résume pas à cette démarche partenariale. Dans le prolongement des réflexions et travaux menés par le passé, je souhaite que nous réformer en profondeur la gouvernance des politiques de protection de l'enfance en nous interrogeant notamment au niveau national sur leur pilotage insuffisant. En dépit de la création du Conseil national de protection de l'enfance en 2016 le regroupement et le renforcement des institutions existantes trop morcelé. J'ai demandé pour ce faire à l'Inspection générale des affaires sociales ne me proposer des scénarios techniques. D'évolution sur ce point j'attends leurs conclusions dans les prochaines semaines, ça aurait dû arriver mais. La crise que nous avons traversée a a très légèrement décalé les choses, mais c'est une priorité, là aussi, ça peut paraître un peu techniques ou techno, mais je pense que c'est assez fondamental dans la conduite de nos politiques publiques de protection de l'enfance, et notamment pour garantir cette égalité. Territoriale que vous évoquiez, madame la la rapporteure. évidemment, cette réforme du pilotage local aura des prolongements et des Rami signifie ramifications territoriale. Les observatoires départementaux de la protection de l'enfance, prévu dans la loi 2007, sauf erreur, ne sont pas encore effectif sur l'ensemble des territoires dans l'ensemble des départements. Les choses avancent, il faut qu'elle s'accélère, là aussi, au niveau local, il faut que le pilotage se renforce avec la pleine participation des enfants là aussi. Cette stratégie, c'est un point important qui me tient à coeur, contient également une exigence très forte d'amélioration de la qualité. Et des contrôles. Des lieux d'accueil des enfants qui doit passer par un renforcement des normes en la matière. Social est un des seuls lieux où il n'y a pas de norme pour les taux d'encadrement par exemple. étonnant. De mon point de vue. Il faut que l'on avance sur ces chantiers-là et le contrôle n'exclut pas la confiance et les Liens qui peuvent être tissés et qui doivent être fort entre les départements et les établissements. Au contraire, je pense que le contrôle est une condition de la confiance. Et tout ça pour le bien de nos enfants. c'est la raison pour laquelle j'ai saisi en janvier dernier, le Conseil national de la protection de l'enfance pour qu'il puisse me faire d'ici le mois d'octobre des propositions d'évolution législative et réglementaire visant à mieux définir les taux d'encadrement des enfants dans les lieux d'accueil. Parallèlement, j'ai demandé à l'ensemble des préfets d'ici l'été, de me faire remonter un état des lieux précis des plans de contrôle des structures existant, c'est dans la loi, qu'en est-il dans les faits. Dans les départements et des démarches conjointes que peuvent mener état et département quand ils sont face à un dysfonctionnement. Enfin, sachez que j'ai saisi l'Inspection générale des affaires sociales, une mission de contrôle, cette fois-ci. Mais aussi pour que nous connaissions davantage la situation précise. Des jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance et qui sont actuellement accueillis, hébergés dans les hôtels. Un drame. Ces produits en janvier dernier. Entre 2 jeunes. Dans un hôtel du département des Hauts-de-Seine. Je veux qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, je veux que ce soit l'occasion pour nous tous, nous ayons d'une part, vous l'évoquiez madame la rapporteure une situation précise. Combien d'enfants dans les hôtels. On ne le sait pas. Ce n'est pas admissible. Et essayer ensemble de trouver des voies de sortie d'amélioration. pour cette situation-là, donc là aussi, l'IGAS été mentionné mais à cet égard-là. Alors vous abordez madame la sénatrice dans notre proposition de loi, le sujet des mineurs non accompagnés des jeunes majeurs, le sujet de la sécurisation des statuts et des parcours des mineurs non accompagnés, notamment la facilitation de leurs conditions de séjour et de travail d'un sujet de vigilance pour moi, évidemment, plus que de vigilance même d'engagement et nous travaillons d'ores et déjà depuis plusieurs mois avec les ministres Christophe Castaner et Muriel Pénicaud, qui confirmé leur leur souhait de faciliter leur parcours en activant de manière prioritaire, les outils de droit commun, parce que moi je. Je crois beaucoup que c'est le droit commun qui doit être mobilisé, plus fortement probablement pour ces jeunes, mais que c'est ça que nous leur devons une fois encore. Je pense notamment au patient à la garantie jeunes. Il y a antigènes antigène sur lequel on sent qu'il y a des dizaines de réflexions peut-être plus large encore en ce moment mais et soyez bien certains, nous faisons en sorte que les jeunes de l'aide sociale enfants soit au coeur des réflexions qui ont cours ou encore au service civique. Faut là encore je pense et je suis sûr que vous en serait sensible partir aussi d'expérience concrète qui ont lieu sur les territoires qu'il s'agit d'identifier et d'évaluer et éventuellement de généraliser, je pense, notamment, en la matière, à ce qui se passe dans le Haut-Rhin, avec des coopérations entre départements, associations, Pôle emploi, les services d'aide à la personne pour favoriser l'emploi des mineurs non accompagnés qui sont devenus majeurs et ça marche. Et ça marche. n'est pas simple des mineurs non accompagnés, je partage avec vous, évidemment la préoccupation fondamentale à l'égard des jeunes sortant à la majorité de l'aide sociale à l'enfance je rappelle que cette attention s'est traduit dès la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit, vous le savez, un volet obligatoire de lutte contre les sorties non accompagnées de l'aide sociale à l'enfance, une fois la majorité atteinte, ce sont 12 millions d'euros qui ont été pour la première année, affecté à louer. Uniquement sur ce sujet à l'ensemble des départements puisque, à une exception près et demi, 2 exceptions près, l'ensemble des départements on contractualisé dans le cas du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, ces 2 millions d'euros qui Servent notamment, et je vous donnerai des chiffre tout à l'heure si vous le souhaitez, plus précis, sert notamment à financer le maintien d'un lien. Ce qu'on sait que le maintien du lien. Et assez cardinal. Mais aussi parfois à financer un complément pour le logement. 12 millions d'euros, donc à cet égard dans la cave du la prévention contre la pauvreté, par ailleurs, sachez, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous expérimentons nationalement avec l'image, un fonds de solvabilisation à destination des jeunes pour les aider à payer leur reste à charge ou pour leur fournir une avance en attendant en attendant je travaille par ailleurs avec Julien Denormandie à affiner les besoins des jeunes sortant de l'aide sociale en France sur les volets logement hébergement, nous savons tous que sur ce volet-là. Créer des droits un droit au logement qui soit opposable ou pas. C'est bien mais ce n'est pas forcément effectif, ce qui compte, c'est de trouver des dispositifs. Qui change véritablement le quotidien de ces jeunes et nous faisons davantage le pari de projets d'expérimentations que nous menons dans les territoires, notamment avec la banque des territoires, c'est un acteur majeur sur ce sujet-là et qui mène, qui, lui, accompagne des projets de résidence sociale qui spécifiquement des jeunes sortant de l'aide sociale en France, en Rhône-Alpes, à Marseille ou encore à La Seyne-sur-Mer. Il faut bien entendu amplifier ces démarches sécuriser la situation de ces jeunes, je vais en autre exemple que nous renforcions vous l'évoquiez madame la rapporteure, la connaissance et la bonne appropriation du dispositif de consignation de l'allocation de rentrée scolaire. Qui a été prévu instaurée vous l'avez rappelé par la loi du 14 mars 2016, porté notamment par Laurence Rossignol, qui a concerné l'année dernière, plus de 47000 enfants ont l'aide sociale confié pardon à l'aide sociale en France, si plus de 3000 jeunes ont récupéré l'année dernière, leur pécule auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Près de 12000 jeunes qui dispose d'un compte non pas depuis la place, la mise en place du dispositif, il y a 4 ans, ils n'ont pas entamé de démarche. C'est de l'argent qui dort. Alors vous avez des jeunes qui en ont besoin, a probablement Donc il faut véritablement que nous renforcions la connaissance de droit, voir ce qu'on peut aller vers une automatisation. L'attribution de ces droits, une fois la majorité, bref c'est des sujets sur lesquels nous avançons et nous travaillons, c'est pas normal que ces droits ne soient pas activé de la sorte, alors qu'ils sont nécessaires à l'adoption. à laquelle est consacré majorité une grande partie des articles votre proposition de loi fait également partie intégrante de la stratégie que nous sommes en train de déployer le rapporteur le le rappelait, c'est d'ailleurs suite aux conclusions d'une enquête menée par l'IGAS sur l'ensemble de la procédure d'adoption dans le département de Seine-Maritime, vous vous en souvenez probablement que j'ai souhaité faire de sur ce sujet, une priorité de mon action, c'est par ailleurs un sublime sujet je dis ça devant votre collègue Imbert, le rapport de l'IGAS, à l'époque que nous, disait-il, d'une part qu'aucun système discriminatoire systématique n'avait été institutionnalisé, c'était la question qui était posée à l'époque et que se pose encore un certain nombre de nos concitoyens dans les fermes, soyons, soyons clairs, mais qu'un ensemble d'usage de pratiques comme les propositions d'enfants couples homo parentaux célibataires ou les demandes d'informations qui était faite pouvait-elle s'avérer discriminatoire, comment n'étions arrivons la cause de procédure d'adoption insuffisamment transparente de modes de désignation et le fonctionnement des conseils de famille parfois trop opaques et d'outils de pilotage par l'état de la politique de l'adoption, une fois encore absent. Il y a nécessité d'ouvrir un peu les portes et les fenêtre s'. Et que la puissance publique reprenne un peu la main de façon très légitime, au niveau national et territorial sur ces procédures. Mais ne méprise action a été d'élaborer une charte de déontologie rappelant certains principes fondamentaux Simple rien nouveau mais c'est mieux en le disant, comme on dit, et qui serait signé par l'ensemble des membres des commissions d'agrément des conseils de famille, elle a été effectivement signé par chaque conseil de famille entre septembre 2000 19 et janvier 2020. Nous ne pouvions évidemment pas nous arrêter là, c'est pourquoi les mesures pour améliorer l'adoption font partie de la stratégie que je défends. Elles font l'objet d'une mission bipartite avec l'Assemblée des départements de France, qui a été conduite par la sénatrice Corinne Imbert, que je salue et que je remercie encore pour son excellent travail et par les députés, Monique Limon. Vous avez raison madame est sénatrice de vouloir agir à à ce sujet, quand on sait, ça a été dit que 50 % des enfants pupilles et qui ne sont pas confier en vue d'adoption ont pourtant un projet d'adoption, mais le conseil de famille n'a pas réussi à leur trouver une famille, on le sait, 14000 familles en France ont eu un agrément

Situation de handicap fratrie, âgés. Qui ne trouvent pas de famille. Il faut donc renforcer l'accompagnement des projets d'adoption et que nous puissions facilité fluidifié ses projets délaissement, suivant ainsi la voie de la ministre signale des sénatrices Meunier Diniz à l'époque et mieux accompagner l'adoption ça vous avez raison sur le l'objectif. Je pense ça ne relève pas forcément de la loi mais plus des pratiques de la formation, l'accompagnement des usages. Les pistes mentionnés sont par exemple sel néanmoins d'un outil national sur l'adoption nationale de référentiels nationaux et de la conciliation de la de la formation de l'ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants et des familles, les procédures d'agrément d'adaptabilité d'accompagnement des parents adoptants doivent être. également davantage précisée sécurisé selon moi et je vous le disais, moi je veux, c'est un. Conviction un combat, je veux que l'on facilite l'adoption des familles, des enfants, pardon à besoins spécifiques, on a fait un déplacement je sais plus Corinne était là mais en tout cas avec Monique Limon, dans le Pas-de-Calais. Il y a 15 ans, le psychologue du service : adoption du Pas-de-Calais a décidé département excusez-moi l'expression se spécialiser. Sur l'adoption des enfants à besoins spécifiques. Et il a monté une méthodologie enfin un discours d'accompagnement des parents. Pour leur expliquer que oui. Même s'ils n'adoptent pas un enfant de 3 mois. En bonne santé mais un enfant plus âgé, éventuellement avec une situation situation de handicap, mais ils seront quand même des vrais parents. Et ça sera quand même leurs vrais enfants. Et ils s'aimeront comme tout parent avec tout enfant. Donc c'est tout un cheminement. Des parents. Vers ce type d'adoption et on a rencontré à l'époque de parents qui avaient s'étaient engagés dans cette démarche-là et qui étaient les plus heureux des parents.

Ces données des parents un enfant et il y a des enfants qui ont besoin de parents voilà et qui aujourd'hui n'en ont pas. Oui, c'est les 2, c'est les 2 et on a eu tendance à considérer que c'était plutôt lent voilà de toute façon en ces matières, tout est question d'équilibre très sensé. J'ai souhaité en parallèle que le Conseil national de la protection de l'enfance, ainsi que le comité national qu'on sait, pardon, comité consultatif national d'éthique, ce sont des lieux de représentation et de concertation, par essence, et qui disposent de l'expertise nécessaire complète par des avis et des recommandations, les propositions des du rapport Limoux Imbert sur l'adoption avant que nous puissions les traduire par des mesures législatives et ses avis m'ont été officiellement respectivement mis remis fin novembre et début mai et nous n'attendons maintenant plus que. Opportunités parlementaire pour pouvoir porter tout cela devant vous voilà ces différents éléments, j'en conclus sont l'occasion pour moi d'inscrire les sujets portée par votre proposition de loi dans la cohérence globale de mon action, nous aurons l'occasion d'échanger, de débats dans le détail sur ces différents articles mais je conclurai en indiquant que certaines des dispositions que vous proposez me semble s'inscrire. De manière pertinente et adaptée aux orientations et travaux que j'ai cités. Et à l'action globale cohérente que je tente de mener. Et que leur insertion conforte l'édifice juridique et législatif qui a été construit jusqu'à présent cependant je l'évoquais à l'instant, cet édifice repose sur un équilibre sensible. Complexe un parce que c'est de l'or de l'intime, tout ça. Voilà. L'intime parfois le président disert. C'est pas forcément la loi qui est en mesure de dire ce qui doit être fait. Ou on pas faire. Et il faut laisser une certaine liberté marge de manoeuvre aux professionnels qui exercent au plus près des réalités. Mais notre boussole commune, c'est la défense des intérêts de l'enfant et la réponse à ces besoins fondamentaux et ne pas s'équilibre ne peut pas être fragilisée par une mise de côté, trop rapide, trop peu automatique de l'environnement familial. De vie de l'enfant, au risque d'aller à l'encontre des droites de ce dernier des droits des parents et c'est là où il faut que nous soyons je pense précautionneux, les uns et les autres, voilà je vis à ce type davantage convaincus que nous avons davantage intérêt à fluidifier accélérer nos procédures, accompagner, former les professionnels, de manière interdisciplinaire et inter-institutionnel qu'à prendre le risque de rigidifier le droit. Au risque de passer à côté d'une évaluation fine nécessaire de chacune des situations voilà Mesdames et messieurs les, les, c'est triste, c'est les sénateurs je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler de ce sujet-là. Et je vous remercie. Merci monsieur le secrétaire d'État. à la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Madame, Esther Benbassa pour le groupe CRCE, vous avez 6 minutes chers collègues. Merci madame la présidente, madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je souhaiterais débuter cette intervention en remerciant les travailleurs de l'aide sociale à l'enfance comme nos médecins, infirmiers et tant d'autres professions elle et il se sont mobilisés pendant la crise sanitaire que traverse notre pays. Ils font actuellement face à la pandémie, avec courage et solidarité et nous leur devons beaucoup. Mes chers collègues, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui elle nous interpelle avec gravité en France 2 enfants meurent chaque semaine un viol sur mineur a lieu toutes les heures, environ 73000 enfants sont victimes de violences, chaque année, et il est à craindre que toutes ces atteintes faites aux jeunes en difficulté, été exacerbée par le confinement. Alors que la protection de l'enfance, devrait être un pilier fondamental de l'égalité des chances, afin que chaque mineur de ce pays puisse s'épanouir et se construire en citoyen modèle notre système reste largement perfectible. Pour cette raison, le texte proposé par notre collègue Josiane Costes, que je salue et les membres du groupe RDSE et bienvenue, pointant du doigt les dysfonctionnements de l'ASE le manque d'investissement de l'État et les lenteurs procédurales contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant Madame Cosse nous présente une proposition de loi intéressante venant apporter certaines réponses aux problèmes majeurs soulevés par le Conseil national de la protection de l'enfance. Jusqu'à présent, le législateur s'est donné pour mission de préserver un équilibre entre le maintien des droits liés à la parentalité et l'intérêt supérieur de l'enfant en a découlé 2 échecs majeurs, tout d'abord l'obstacle à l'adoption, qui empêche actuellement à des personnes le souhaitant d'accueillir aisément un enfant dans leur foyer, deuxièmement des procédures de délaissement longue et fastidieuse qui plonge certains mineurs dans des situations de précarité avec des parents souvent violents ou incapables de les élever. Trop longtemps, le législateur est parti du postulat que les Liens du sang devait primer et l'enfant se maintenir le plus longtemps possible dans sa famille biologique. Ces traditions devrait impérativement prendre fin oui, certains parents ne sont pas aptes à élever leurs enfants, oui, ces enfants doivent être mis à l'abri, protéger et confiés à des familles adoptives qui sont susceptibles de réunir les conditions essentielles à leur épanouissement ainsi les auteurs de ce texte ont souhaité rendent le recours à l'adoption. Simple à l'adoption La filiation par adoption simple n'effaçant pas la filiation biologique, les tuteurs adoptive prendront le relais des parents de sang pour les 2 l'éducation des enfants délaissés Le dernier pan intéressant de ce texte et le traitement qui est fait des mineurs étrangers alors que le gouvernement continue à fermer les yeux sur leur enfermement ensemble de rétention administrative, au détriment des préconisations de la Cour européenne des droits de l'homme, cette proposition de loi nous rappelle un élément fondamental avant d'être des étrangers, ces mineurs sont des enfants. Qu'il faut éduquer intégré et surtout protéger en permettant à ces derniers d'accéder plus aisément à un type de séjour en simplifiant les règles d'adoption pour les enfants nés à l'étranger, ce serait de véritables pas fait pour la normalisation de leur situation, si ces mesures ont été adoptées nous change Lyon de paradigme l'enfant primerait sur le migrant. De tels éléments viserait à rendre plus humaine, nos politiques d'accueil des mineurs étrangers et nous ne le salut à Lyon que positivement ces évolutions cependant certaines dispositions proposées dans ce texte semble éloignée des réalités de terrain voir compte productive, c'est notamment le cas des conditions de reprise des enfants placés posé à l'article IV. Pour cette raison le groupe CRCE s'abstiendra sur cette proposition des lots de loi nous sommes cependant favorable à ce que des travaux soient menés sur une telle sujet c'était d'ailleurs le sens de notre proposition de loi visant à créer une délégation parlementaire aux droits des enfants rejetés par notre assemblée, le 20 novembre 2019, mes chers collègues, nos enfants sont l'avenir de notre pays, actuellement 300000 mineurs sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, eux aussi ont le droit à un avenir meilleur, a une citoyenneté épanouissante a insulté économique et à un accès sécurisé à l'éducation et à la vie active Sims nous menons ce combat de front leur futur n'en sera que plus stable et enviable, je vous en remercie, merci. La parole est maintenant à Madame Élisabeth Doineau, pour l'Union centriste, si vous avez 8 minutes. ça me la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, chers collègues, c'est vraiment un grand plaisir de rejoindre cet hémicycle en tout cas pour cette merveilleuse occasion cher Josiane Costes pour parler de la protection de l'enfance et je vous en remets. Une fois n'est pas coutume effectivement que nous abordions ce sujet et, en réalité, ce sujet devrait sortir de cet hémicycle, bien plus souvent parce que la réalité dans nos départements, c'est que c'est un sujet alors c'est d'actualité confinés, en réalité, personne n'a envie de parler de la protection de l'enfance parce que c'est une défaite que des enfants soient abandonnés, c'est une défaite que des enfants soient et en réalité c'est toujours caché et je crois qu'aujourd'hui, nous en parlons ici mais surtout demain, parlons-en dehors et par le 11 ans avec vraiment beaucoup de fièvre et d'envie de travailler tous ensemble il est louable de sortir des rapports de sortir, voilà des écrits de dire beaucoup de choses sur la protection de l'enfance, mais je crois surtout, il faut mettre notre énergie dans l'action. La réalité c'est que la protection de l'enfance, ça reste effectivement un sujet tabou, il faut sortir de ce tabou parce que ces enfants-là sont aussi nos enfants, ce sont aussi des enfants de la France et nous ne devons pas les oublier, une fois n'est pas coutume nous parlons donc de la protection de l'enfance, une fois n'est pas coutume et je voudrais remercier le cabinet du ministre parce que pendant toute la période de l'de la pandémie en tout cas, en charge de la protection de l'enfance dans mon département, j'ai pu remarquer combien vous étiez mobiliser les uns et les autres alors c'est toujours un peu trop tard, c'est toujours un protocole, un peu trop long qui nous arrive, mais en réalité on a pu voir votre énergie à à répondre à nos attentes et surtout à enregistrer nos questions parce que nous avions beaucoup de questions sur le terrain et vous y avez toujours répondu avec beaucoup de précision et la plus grande célérité, je crois que vous pouviez avoir donc, merci monsieur le ministre, et merci à ceux qui sont à vos côtés qui représente toute votre équipe moi je voudrais aussi me joindre remerciements qu'a fait Esther Benbassa tout à l'heure pour tous les acteurs de la protection de l'enfance, il y a effectivement tous ces professionnels médecins agents tout simplement du conseil départemental, les, comment les éducateurs, bien sûr, mais tout ce qui gravite autour de la protection de l'enfance, et en particulier les assistants familiaux parce que les assistants familiaux, ne l'oublions pas, ils ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 2 mois et demi et il mérite effectivement que nous ayons beaucoup de reconnaissance, ils sont aujourd'hui épuisées les assistants familiaux, j'espère que les départements seront tous mobilisés pour leur accorder ce qu'ils leur doivent pour avoir accueilli ces enfants et les avoir accompagné sans le soutien pour les enfants, par exemple, qui était avec des problématiques de handicap, hé bien 2ème ou des ITEP qui malheureusement était fermé et donc je peux vous assurer que, aujourd'hui, nous devons avoir cette reconnaissance et, plus encore, c'était une une astreinte très longue, je pense que nous devrons d'ailleurs réfléchir au statut des assistants familiaux, Monsieur le Ministre, parce que il y a certainement à la marge quelques avancées à à faire sur ce sujet, en réalité, leur statut n'a pas beaucoup bougé depuis des années et on voit que le monde bouge, que les enfants sont de plus en plus complexe, enfin, ont des profils de plus en plus complexes et je crois que nous devons réfléchir à leur profession alors moi ce que je voulais dire, je voulais sortir finalement chers collègues de de votre texte que que j'ai trouvé très ambitieux, c'est, c'est c'est sans doute très bien d'être ambitieux et et je pense que il y a une multitude de sujets dans votre texte, on n'a pas l'habitude ici, traiter des PPL avec autant d'articles, c'est vrai que c'est souvent des pupilles, elle a un article unique et et quelques fois sans doute ça frustre, alors là, nous n'étions pas frustrée parce que nous avions tous les six, c'est-à-dire que lègue à vrai dire, moi ça fait 15 ans que je suis engagé dans la protection de l'enfance dans mon département et et donc j'ai cherché un comme raccrocher dans vos dans je me suis accroché effectivement à tous les sujets, ils sont tous intéressants, je pense que il est effectivement il y a des des travaux à mener, mais pour autant, c'est vrai que j'ai, j'ai un petit peu eu du mal, j'étais troublé par les propositions des articles et et je vous prie de cette cette spontanéité que j'ai envers vous mais j'ai été troublé en quelque sorte, parce que je ne me suis pas reconnu dans ces problématiques dans mon département, réalité mais je, je veux bien travailler avec vous sur sur tous ces sujets, moi je pense qu'il y a 3 difficultés aujourd'hui dans la protection de l'enfance, le 1er c'est que la protection de l'enfance n'a jamais été financée à son juste niveau, c'est-à-dire que c'était une décentralisation à l'époque, certes bienvenue mais je pense que là, on peut parler de délaissement on a délaissé au département cette responsabilité sans leur donner le moindre sou et c'est ça l'erreur, c'est ça l'erreur parce que c'était en réalité une mission essentielle pour les départements le 1er problème c'est le financement parce que le Fonds national de protection de l'enfance n'a jamais été abondé à son juste niveau et je remercie le ministre aujourd'hui d'avoir, comment organiser, c'est cette stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance parce que là, du coup, effectivement, ça nous a permis de réfléchir tous ensemble sur les sujets les plus importants de travailler le fond et j'ai trouvé votre méthode excellente, monsieur le Ministre, alors moi je ne suis pas la République en marche alors vous m'excuserez mais je quand il y a des compliments faire je l'ai fait et la réalité, c'est que j'ai beaucoup apprécié cette méthode et et donc de concertation et que la contractualisation avec les départements, hé bien c'est quelque chose qui va aussi apporter beaucoup en qualité et surtout ça ça permet d'avoir aussi des financements pour la première fois en fait, en réalité, la protection de l'enfance aura des financements en en échange effectivement d'une certaine qualité de pratiques et d'innovations, et c'est là justement le 2ème point que je voulais aborder après le financement, le 2ème point c'est effectivement la problématique de faire changer, de faire bouger les lignes dans nos équipes départementales

qui l'avait important pour nous dans notre département, d'avoir eu une inspection de l'IGAS pendant quelques mois pour justement amener les professionnels à réfléchir sur leurs méthodes et sur les changements de leurs méthodes et surtout de leur approche et donc moi ce que je suggère au gouvernement c'est de mettre en place des équipes qui irait dans les départements qui ne serait pas seulement sur le contrôle et surtout pas sur le contrôle, mais sur cette espèce d'énergie de dynamique à créer sur l'innovation et sur la recherche d'autres méthodes et je pense que ces petites équipes qui passerait passerait dans les départements pourraient justement aller très très vite vers une amélioration de ce qui ne se fait pas bien dans certains et en tout cas, ça permet aussi de diffuser les pratiques de ce qu'ils font très bien dans les départements, le 3ème point que je voulais aborder, c'est elle, les relations tuyaux d'orgue aussi que malheureusement nous vivons quotidiennement entre les départements, la PJJ et les services par exemple de la santé et notamment de la psychiatrie, ça, c'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrive à se comprendre entre la justice et la protection de l'enfance, il faut qu'on arrive à se parler aussi avec avec la pédopsychiatrie, en réalité, vous voyez, il y a, il y a 3 chantiers, le financement, vous l'avez commencé avec la stratégie, il le confie à nos plein ah oui pardon, j'ai pas vu que j'ai dépassé mon temps, enfin voilà, je voulais vous dire tout mon enthousiasme, parler de la protection de l'enfance, de l'enfance, alors merci, cher collègue et merci au ministre d'aller encore plus loin dans dans la qualité des pratiques merci. Merci, et merci de respecter votre temps. La parole est maintenant à Madame Nicole Duranton pour le groupe Les République. Qui a osé 4 minutes merci madame la présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, le nombre de mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance est en 2020, estimé à 350000 contre 300000 en 2017, 2017, 7 E O s'explique par une meilleure détection des cas critiques, par le biais des enseignants et des assistants sociaux, dans les familles, mais c'est aussi le constat d'une situation de plus en plus inquiétante avec le confinement dus à l'épidémie du Covid 19 les violences intrafamiliales ont augmenté et en particulier la la maltraitance à l'égard des plus jeunes, la protection de l'enfance et l'un des aspects cruciaux de la politique d'égalité des chances, en France, elle vise en effet à offrir une prise en charge, garanti par l'État, partout où l'autorité parentale est défaillante, la prise en charge est loin d'être parfaite, même si je tiens à féliciter les personnels de l'ASE qui font beaucoup avec peu, ainsi que tous les professionnels impliqués services départementaux association magistrats et les familles d'accueil recevant ces jeunes, je prends l'exemple de mon département, dans l'Eure en 2015 le nombre d'enfants placés, il était de 1845 en janvier 2020, ce chiffre est de 2300 453 assistants familiaux, travaille pour le département, ces familles accueillent plus de 60 % des enfants placés les 40 % restants se répartissent en six maisons d'enfants à caractère social 15 lieux de vie et d'accueil et un foyer de vie et de l'enfance pour toutes ces structures, le budget de l'ASE dans l'Eure et de 70 millions d'euros pour l'année 2020, l'État a un triple rôle piloter la politique de l'Enfance contrôler la qualité des dispositifs et créer du partenariat avec les conseils départementaux en effet 80 millions d'euros ont été débloqués en octobre dernier et c'est une bonne nouvelle pour la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance et leur fait partie des 30 départements sélectionnés pour en bénéficier, en co-finançant les projets du département, l'objectif est de donner aux jeunes placés les mêmes chances qu'aux autres, les critiques se multiplient contre les foyers et les structures d'accueil de ces mineurs il y a des délais importants 31 % des pupilles de la nation sont admis après une prise en charge de 5 ans, il s'agit ainsi de repenser la durée des procédures et de mieux gérer chaque parcours et je salue la volonté de mes collègues RDSE notamment Madame Coste de revoir cette question complexe sans faux-semblants, tout le monde veut bien faire, car la protection de l'enfance est une tâche noble cependant cette proposition de loi fait de l'intérêt de l'enfant, le seul marqueur unique et absolu de cette politique, or les besoins médicaux sociaux les modes de garde l'intérêt des parents et de la fratrie doivent être aussi pris en compte la vie de l'enfant n'est pas exemple des de revirements, ce sont tous ces besoins complexes et parfois opposées que la loi doit synthétiser cette proposition de loi semble employer un raisonnement quelque peu paradoxale : d'un côté, elle s'appuie sur le désir de parentalité, or être parent n'est pas un droit, c'est un devoir, et même une série de devoirs d'un autre côté, elle envisage notamment dans ses articles 3 et 4 un recours prioritaire à l'adoption le plus tôt possible lorsque cette parentalité est défaillante, arguant du fait qu'un enfant pourra ensuite explorer s'parente biologique, alors même que l'on sait pertinemment que l'adoption est complexe et parfois traumatisantes, la responsabilité des mineurs revient légalement à leurs parents, l'autorité parentale, cette valeur chère à notre famille politique doit rester au coeur de la décision, l'État doit intervenir lorsque c'est nécessaire, en particulier durant cette période de crise sanitaire, mais en aucun cas déresponsabiliser ou se substituer aux parents, ce sujet est encore trop souvent tabou, l'ambition de tous et d'éveiller la conscience collective quant aux violences subies par les enfants, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Sueur. Vous avez 5 minutes sur président. Merci madame la la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci à Josiane Costes, de nous avoir conduit à traiter de ce sujet si important. Parce que il y a la convention internationale des droits de l'enfant. Que la France a signé mais. Combien de lignes de ce texte reste des lignes morte et non respecté, donc il y a aujourd'hui, chiffres 2018 306000 mineurs pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, les juges pour enfants ont été saisis en 2018 de 126145 mineurs en danger 122 mineurs ont été victimes d'infanticides en 2018. Les nombreux d'appels au 119 numéro d'urgence pour l'enfance en danger, ont augmenté de 113 % pendant les 2 mois du confinement, la plateforme en France, danger, a vu les appels, augmenté de 56 % par rapport à l'an dernier et face à cela, Monsieur le Ministre, vous le savez, il y a un grand travail, cela a été dit, de l'ensemble des personnels de l'ASE dans tous les départements de notre pays, il y a des enfants victimes de violence, et à cet égard je dois au nom de notre collègue, Madame Michelle Meunier regretté que 2 amendements qu'elle avait déposé été retoquée une fois encore, en vertu du fameux article 45 de la Constitution qui est toujours appliquée ici dans des conditions que je juge déplorable, car enfin, on peut dire que ça va de soi, ça va de soi que l'éducation que l'action sociale ne doivent s'exercer afin qu'aucune violence morale ni physique, ça va de soi, mais il est peut-être il est en tout cas, c'est ce qu'a pensé madame Michelle Meunier qui m'a chargé de vous faire part de sa réaction, s'agissant des articles 1 2 et 4 nous partageons totalement la position de monsieur Alain Marc notre rapporteur, car nous pensons que ces mesures pourraient être préjudiciables à l'enfance au lien entre les parents et les enfants à la possibilité qui doit être donnée aux enfants : oui aux parents et suis chez moi de revenir en arrière par rapport à un certain nombre de procédures. Pour ce qui est des allocations familiales, nous avons proposé un amendement de suppression de l'article 9. Pour laisser une capacité d'appréciation au juge qui nous paraît être finalement une bonne chose et je remercie la commission, monsieur le président d'avoir elle aussi repris cet amendement, je terminerai par quelques mots sur les mineurs isolés non accompagnés, monsieur le ministre, d'abord je voudrais redire mais vous l'avez entendu si souvent, vous en êtes persuadé qu'il faut un plus juste équilibre sur le plan financier entre l'État et les départements pour la prise en charge des mineurs non accompagnés, c'est une nécessité aujourd'hui les départements ne pourront plus continuer à assumer cette mission dans ces conditions. Ce que propose Madame Cosse c'est très intéressant, introduire une présomption de désintérêt pour faciliter la prise en charge de ces jeunes par les services de l'enfance désigné le juge des enfants pour ces mineurs encore qu'on puisse en discuter en effet favoriser l'accès à un compte en banque, lorsque des mineurs reçoivent une bourse et que ils ne peuvent pas l'apercevoir, il y a quand même, qu'est que, chose qui ne va pas et notre collègue Jean-Yves Leconte présentera un amendement très précieux à ce sujet, tout à l'heure, favoriser l'attribution de titres de séjour au bénéfice de mineurs non accompagnés, intégré dans un cursus professionnel enfin généralisé, l'accompagnement des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans, ce sont Madame Coste, des mesures qui vont dans le bon sens, c'est 40000 jeunes en effet, cela a été dit précédemment, c'est d'abord des être s'humains, ils sont là. Ils sont là, et vous savez, mes chers collègues, que seulement 42 % de ces personnes de ces jeunes sont reconnus mineurs alors les autres, madame la présidente, il doit faire un recours, c'est très compliqué et ça pose des quantités de problèmes donc ce sujet, il est encore largement devant nous et merci à la faveur de cette proposition de loi de savoir donner l'occasion de l'évoquer ici, je sais que vous entendrez ce message, monsieur le ministre. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Xavier il y Covili pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi relative aux mineurs vulnérables dans un contexte de crise sanitaire qui frappe en 1er lieu les publics les plus fragiles, cette proposition de loi couvre à travers 15 articles on le rappeler 15 articles c'est une PPL chargé. Un Champ très large et traite des problématiques aussi diverses que complexes, je voudrais commencer par saluer la démarche de l'auteur, notre collègue Josiane Costes pour la proposition de cette loi qui permet d'évoquer des sujets essentiels tels que l'adoption, la protection de l'enfance, l'accompagnement des jeunes majeurs et des mineurs isolés étrangers, elle permet de mettre en lumière une fois de plus, un certain nombre de problématiques et de dysfonctionnements auxquels nous devons apporter des solutions concrètes dans l'intérêt des enfants et des jeunes vulnérables, elle s'inscrit également dans un contexte global dans lequel l'ensemble des acteurs sont mobilisés, le Parlement s'est souvent investi de cette question, je pense au rapport de la députée Perrine Goulet au rapport de la députée limon et de notre collègue Imbert sur l'adoption et sur la PPL que j'ai déposé en juillet dernier avec notre collègue Nassima Dindar et dont plusieurs de notre collègue sur tous les bancs ont cosigné cette PPL qui traiter un certain nombre de sujets dont celui de la prise en charge des jeunes majeurs, le gouvernement par votre voix, monsieur le ministre est également mobilisés dans le cadre de la stratégie nationale pour la protection de l'enfance 2020, 2000 22 et qui aboutira nous l'espérons, à de réelles avancées en matière de protection et d'accompagnement, enfin, on constate une prise de conscience collective partout dans la société grâce en 1er lieu aux enfants placés qui ont largement contribué à libérer la parole et qui chaque jour nous rappelle qu'il est urgent d'agir, les 3 axes de cette PPL, à savoir le délaissement parental l'adoption, la prise en charge des jeunes majeurs et la protection des mineurs isolés étrangers constituent des problématiques complexes mais bien réelle dans l'ensemble du territoire en ce qui concerne la le délaissement parental, l'article 2 supprime la proposition de mesures de soutien aux parents des laissant nous partageons l'objectif de cette disposition qui vise à placer l'intérêt supérieur de l'enfant en haut des priorités mais nous pensons qu'elle crée un déséquilibre au regard de la nécessité des mesures de soutien à la parentalité, notamment avec un délai trop restreint, celles-ci ont notamment montré leurs vertus du grand confinement, période où les tensions peuvent être plus importantes, notamment chez les familles les plus précaires vivant dans des espaces restreints. Nous croyons donc à la nécessité de trouver un juste équilibre en protégeant en 1er lieu les enfants et en accompagnement davantage on accompagnant davantage les parents en difficulté, telle est l'objectif du gouvernement, tant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance que j'évoquais, mais également Monsieur le Ministre, avec le programme des 1000 premiers jours de l'enfant que vous avez mis en place dernièrement, accélérer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental pourraient également ça inefficace, notamment au regard du fonctionnement de la justice et de la délicate appréciation du délaissement parental sur l'accompagnement des jeunes majeurs et la problématique des sorties sèches, je le dis, personne ne peut accepter que la rue, à 18 ans, soit la seule option pour ces jeunes aujourd'hui, rappelons-le, 70 % des jeunes de la ASE sortent sans diplôme 40 % des personnes sans domicile fixe de moins de 25 ans, on eut un parcours à l'aide sociale à l'enfance 40 % chers collègues, alors même qu'ils ne représentent que 2 à 3 % de la population globale, comment pouvons-nous demander un jeune dans le parcours de vie a été si difficile de faire ses valises, le jour de ses 18 ans alors même que, selon l'Insee, l'âge moyen de décohabitation en France est à 27 ans, ils ont également le droit d'être des Tanguy comme tous nos enfants, le gouvernement a d'ailleurs interdit les sorties sèches durant la durée du confinement et on peut que s'en satisfaire, ce qui va, ce qui est évidemment nécessaire au regard des risques auxquels les jeunes sous protection sont exposés et on pourra en parler dans le débat, dans un dans un certain nombre de départements, des gymnases réquisitionnés pour accueillir les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des gymnases où ils étaient entassés non plus de solution hôtelière, même si pour avoir aussi le débat et solutions hôtelière pour les mineurs ne sont pas forcément la panacée, mais il y a un vrai problème aujourd'hui de prise en charge par les départements. Monsieur le Ministre vous avez récemment transmis une circulaire précisant à la fois les objectifs, le calendrier et les financements des conventions qui seront signés dans d'ici d'ici quelques jours entre les ARS, le préfet, les préfets et les 30 départements volontaires pour mettre en oeuvre et la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, annoncé le 14 octobre dernier la fin des sorties sèches, il est préconisé et nous nous en réjouissons nous saluons la proposition de l'auteur de la PPL visant à rehausser à 3 ans l'âge jusqu'auquel la situation des enfants confiés à l'ASE est examiné tous les 6 mois par la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnel, nous voterons donc pour cet amendement. Il nous paraît en effet essentiel qu'un suivi régulier lieu pour le développement et le Cadre de vie de l'enfant, enfin sur le principe de présomption d'impossibilité d'exercer toute ou partie de l'autorité parentale pour les parents des mineurs isolés étrangers moi je comprends l'objectif visant à déléguer totalement ou partiellement l'exercice de cette autorité parentale, les structures accueillant des enfants se retrouvent en effet confronté à un certain nombre de situations qui dans la vie quotidienne de l'enfant nécessite l'accord explicite des parents parfois injoignable et souvent absent ces barrières juridiques qui empêchent par exemple l'enfant de se rendre à un anniversaire d'un camarade, le week-end, comme tous les autres enfants les prive d'une vie normale et portent préjudice à la sociabilisation toutefois cette problématique concerne les mineurs isolés étrangers mais également tous les publics, prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance, nous devons donc en débattre en concertation avec l'ensemble des acteurs pour trouver sur les actes usuels et non usuels, eu un juste équilibre entre l'intérêt de l'enfant et le respect de l'autorité parentale des parents dans l'application des dispositions en vigueur pour conclure, je voudrais une fois de plus saluer le travail de l'auteur de cette proposition de loi qui pose un débat essentiel mais qui nécessiterait une approche plus globale au vu de l'importance des sujets nombreux évoqué dans cette PPL je vous remercie. Si un collègue, la parole est maintenant Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Merci madame la présidente, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, merci, merci à nos collègues de gauche de faire la démonstration, une fois de plus, de leur obsession alors qu'il prépare une proposition de loi tout ce qu'il y a d'intelligent que tout le monde devrait pouvoir signer dès demain concernant la protection de l'enfance, voilà qu'se débrouille encore pour essayer de nous faire passer la pilule de l'immigration massive, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, si vous faites une loi pour les petits Français, vous vous sentez obligé de faire une loi pour les immigrés en période de crise sanitaire alors qu'une crise économique sans précédent va nous tomber dessus, que des millions de Français vont peut-être se retrouver au chômage et qui sait à la rue avec leurs enfants, vous n'avez qu'une seule priorité : les autres encore les autres toujours les autres, ça c'est pour la logique délirante de votre proposition mais venons-en au fond qui est tout aussi dingue, on dirait que vous envoyez un message à l'Afrique Continents économiquement sinistrées, où la démographie explose, dont environ 40 % des habitants en moins de 15 ans, vous êtes en train d'expliquer à 500 millions de jeunes Africains que s'ils viennent illégalement chez nous, ils seront accueillis à bras ouverts et que la France pourvoira à tous leurs besoins, on le sait, cela a été rapporté ici dans cet hémicycle les fameux mineurs isolés seraient plus de 70 % être en réalité majeur mais comme la gauche et la droite ont refusé de rendre obligatoire les tests osseux, on reste dans le flou : cachez ces clandestins que vous ne sauriez hé bien hé bien ces mineurs isolés, selon votre article 6, ils pourront être pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance jusqu'à leurs 21 ans, c'est-à-dire que l'étranger entre 18 et 21 ans pourra faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais en même temps être pris en charge par l'ASE, c'est-à-dire par les départements et d'ailleurs pourquoi 21 ans, pourquoi pas 22 jusqu'à 30 ou 40, vous allez en plus dévoyé avec l'article 11 le principe même de la nationalité française, puisqu'en cas d'adoption simple simple dire quand l'enfant conserve les Liens avec sa famille biologique, il sera quand même naturalisé français, l'article 15 est un exemple de laxisme le plus total, alors qu'aujourd'hui, pour obtenir une carte de séjour à titre exceptionnel les mineurs non accompagnés, doivent être dans une formation professionnalisante depuis au moins 6 mois, vous voulez supprimer le caractère exceptionnel et que la carte soit des livrables dès le jour où il entre en formation, en résumé, d'abord vous attirer sur les routes de la mort en Méditerranée, des centaines de milliers de personnes qui viendront bénéficier de notre système social, ensuite vous mettez tout en oeuvre ou pour qu'il puisse rester ici toute leur vie, enfin vous allez créer de toutes pièces et des Français, avec ceux qui seront arrivés ici et qui parviendront à se faire adopter, non seulement vous porterez une lourde responsabilité dans les morts qu'il y aura en Méditerranée, mais en plus vous allez encore déstabiliser notre sentiment national, comment être une nation si n'importe qui peut devenir français en un claquement de doigts, votre proposition est délirante mais en plus ça les sournoise et malsaine vous n'assumez pas vos convictions, vous vous cachez derrière la protection de l'enfance à laquelle nous sommes tous attachés, votre votre volonté profonde submerger notre pays de tsunami migratoire que vous transformerez en français de papier autre obsession et là, la disparition de l'identité de la France, merci madame la présidente. La parole est maintenant Monsieur Michel Amiel, vous avez 6 minutes. madame la présidente, pardon, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par Josiane Costes vise à apporter des améliorations aux dispositifs en faveur des mineurs vulnérables sur le territoire national et il faut l'en remercier, ce texte est une Pierre supplémentaire à l'édifice constitué, il faut le dire, d'un amoncellement de rapport en la matière, issu de l'IGAS du CCNE du Parlement, et sans oublier les 2 grandes lois de 2007 et de 2016, tous ces textes visant à la mise en place d'une stratégie pour la protection de l'enfance, si cette proposition de loi et des chances, généreuse, nous restons dans l'expectative d'une réforme globale et de grande ampleur d'ailleurs esquissé, monsieur le Ministre, par vous-même, au nom du gouvernement rendre plus facile l'adoption simple des enfants délaissés, est une idée certes intéressantes, on peut même se demander si elle va assez loin et s'il ne faudrait pas favoriser purement et simplement l'adoption plénière, il est vrai que notre culture juridique de la famille donne priorité à la famille biologique, parfois d'ailleurs au détriment de l'intérêt de l'enfant. C'est pour moi l'occasion de rappeler que l'adoption doit se situer avant tout du côté de l'enfant et que le droit à l'enfant ne saurait se substituer aux droits de l'enfant, quelle que soit sa forme, l'adoption doit rester une modalité de la protection de l'enfance si tout enfant a droit à une famille tout adulte n'a pas forcément droit à un enfant, il y a aujourd'hui en France, beaucoup d'enfants adoptables qui demeure au trop longtemps sans famille et nous ne pourrons échapper à une approche globale, comme vous l'avez d'ailleurs dit Monsieur le Ministre de l'adoption, qu'elle soit simple ou plénière à l'international ou de pupilles de l'État. Concernant la prise en charge des jeunes majeurs au-delà de 18 ans afin d'éviter une sortie sèche de l'ASE comme on dit si elle est une nécessité absolue, elle doit, selon moi, faire l'objet d'un dispositif original sous forme de bourses par exemple car pour beaucoup de jeunes s'émanciper de l'ASE constituent une volonté absolue que l'on peut comprendre si l'on considère certaines parcours particulièrement chaotique. De plus, il existe une grande inégalité territoriale d'un département à l'autre pour des raisons idéologiques et où bien souvent surtout de moyens, raison pour laquelle je plaide pour un pilotage national du dispositif, et pas seulement d'un point de vue observationnelle. à propos des mineurs non accompagnés, rappelons que si juridiquement, ils dépendent aussi du droit des étrangers, ils sont avant tout, avant tout, éligibles au dispositif de protection de l'enfance qui n'exige pas de conditions de nationalité, conformément à la convention internationale des droits de l'enfant que la France a signé et ratifié à ce titre ils dépendent donc des départements et force est de constater, là encore une grande hétérogénéité, raison supplémentaire aux pour moi d'être en faveur d'un dispositif national, même si depuis 2013, un protocole a été élaboré entre l'état et l'association des départements de France pourra instaurer en quelque sorte une double solidarité de l'État envers les départements par un appui logistique et financier lors de l'évaluation du mineur et a entre les départements, par un mécanisme de péréquation géographique afin d'équilibrer le nombre de MNA accueilli qui ne paraît pas forcément très satisfaisant. Pour terminer, je voudrais insister ce qui me paraît de loin le plus important, en citant le préambule de l'ordonnance du 2 février 45. Il est peu de problèmes aussi importants que ce qui concerne la protection de l'enfance, la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elles aient le droit de négliger tout ce qui peut-on faire des être s'. Je défends donc avec force l'idée que la jeunesse est une priorité, et au-delà des mots, qu'elle le doit relever d'une compétence régalienne de l'État régalienne de l'État alors qu'à ce jour, elle se répartit entre la de jeunesse en danger de l'ASE rattaché au ministère des Affaires sociales, la jeunesse réputée dangereuse, confiée à la PJ et donc au ministère de la justice recentré, d'ailleurs, depuis 2007 sur le pénal, ce qui me paraît être une funeste erreur et la jeunesse supposé sans problèmes relevant elle de l'Éducation nationale, alors sous le vent, souvenons-nous de la fragilité de l'enfance, et pas seulement dans ses premières années que naît en considérée comme normale peut basculer à tout moment et que si un enfant en danger peut devenir dangereux, un enfant dangereux, lui, est toujours en danger. Insistons encore et toujours sur l'importance de la prévention dans le domaine sanitaire par exemple troubles psychiatriques madame doit nous la rappeler un trouble psychiatrique de l'enfant dépister précocement peut guérir mais prévention aussi dans le domaine familial et social, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant Madame Françoise Laborde pour 7 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, ces dernières années, le législateur s'est régulièrement emparé de la cause des enfants à la fois sous l'influence d'une prise de conscience au niveau national, de l'impact des violences intrafamiliales dont certains enfants sont victimes d'un contexte international dramatique de guerre et de crise économique, qui jette sur les routes et sur les mers, des familles, leurs enfants et des jeunes seuls pour venir frapper aux portes de l'Europe, mais aussi d'un mouvement juridiques majeurs intervenus au niveau international, bien sûr, des glissements sociétaux ont préparé ce changement de paradigme en France et dans le monde, comme avec la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 contraignante qui a consacré le changement de regard des adultes sur les enfants et qui produit des jurisprudences dont nous ne mesurons pas encore toute la portée, ou encore avec des initiatives non contraignante, comme la déclaration de Genève de 1924 ou la création de l'UNICEF en 1947 ces dernières années, les occasions législative de rendre les droits des enfants plus effectif se sont multipliés de façon transpartisane je pense bien sûr à la loi 2016 sous le précédent quinquennat comme cela a déjà été rappelé et plus récemment à l'adoption de la loi sur les violences éducatives ordinaires ou de celle sur les violences au sein de la famille, ces initiatives ont permis de rendre visible la vulnérabilité de certains mineurs du fait de relations familiales toxiques trop fragile ou inexistante, vous connaissez aussi mon engagement pour la lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs et contre l'inceste dans un 1er temps la médiatisation de ces violences, a permis de sensibiliser la population et de lever les tabous dans toutes les institutions familiales scolaire et même ecclésiastique dorénavant la problématique se déplace vers la question de la prise en charge des mineurs vulnérables, ces derniers mois plusieurs reportages ont mis en lumière les limites de notre système de protection de l'enfance et l'insécurité qui peut à la fois découlait du manque d'encadrement et de l'instabilité des parcours pour ces jeunes, c'est dans ce contexte que notre collègue Josiane Costes, forte de son expérience de conseillère départementale et d'enseignante a décidé de s'engager pleinement devant le Sénat pour porter sa proposition de loi soutenue par mon groupe du RDSE, très soucieuses d'améliorer la protection des mineurs, elle a voulu mettre toutes ses convictions à leur service afin de leur donner un cadre de vie décent, en particulier pour les plus vulnérables d'entre eux, c'est un sujet qu'elle porte depuis de nombreuses années et je tiens à lui rendre hommage pour cette initiative parlementaire, qui ne se contente pas de dénoncer les limites du système de protection de l'enfance actuel, elle propose d'y apporter des solutions destinées à tous les mineurs vulnérables, français et étrangers, je ne ferai aucun commentaire sur ce qu'on a entendu précédemment, d'ailleurs je n'ai pas tout entendu car je me suis boucher les oreilles, je reviens donc à mon texte, ces enfants placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, ces propositions repose sur le constat de l'affaiblissement budgétaire des départements qui est malheureusement une tendance structurelle cet affaiblissement est liée en partie à la performance croissante de la détection des cas problématiques, notamment depuis la loi de 2016, mieux on détecte les cas de maltraitance et plus nombreux sont les enfants à prendre en charge, c'est inévitable, c'est mathématique. Mais surtout la difficulté financière des départements est liée à l'agréable à l'aggravation de la situation sociale sur notre sol au renforcement des inégalités, il y a l'émergence de nouveaux publics, des services sociaux, les personnes admises à l'asile et les mineurs non accompagnés, sans un effort financier supplémentaire substantielle de l'État, il y a crainte que la qualité de la prise en charge des mineurs pâtissent de la dégradation de la situation financière des conseils départementaux dans son travail, notre collègue s'est attaché à adopter une philosophie positive et à poursuivent les travaux dans la direction de la loi de 2016 qui avait, en particulier réformer l'adoption simple de l'art en la rendant irrévocable durant la minorité toutes les propositions de ce texte vise en réalité à ce que l'enfant puisse bénéficier d'une plus grande stabilité d'un accueil dans la dignité et le respect de ses droits, rendant possible un accès à l'éducation, sans être ballottée entre sa famille biologique, les foyers et les familles d'accueil, mais tout en préservant son droit à connaître ses origines, il s'agit de s'élever au-dessus des oppositions classiques de la protection de l'enfance d'une part entre la préservation absolue des Liens biologiques et d'autre part l'idéalisation d'une protection étatique étatique et ainsi de sortir de tout dogmatisme, ce qui est un souci constant des membres du groupe RDSE, comme vous le savez, on confond trop souvent encore l'intérêt supérieur de l'enfant et celui de ses parents, de façon indirecte, ses nombreuses propositions pourraient permettent de repenser l'action des départements au moment où la prise en charge des jeunes Man majeurs et des mineurs isolés étrangers bute essentiellement sur la question financière, comme l'a montré récemment l'examen de la proposition de loi bourguignon à l'Assemblée nationale, rappelons qu'en 2019, selon les chiffres de l'ADF, la seule prise en charge des mineurs isolés étrangers s'est élevé à 2 milliards d'euros, c'est pourquoi il est apparu nécessaire que ces propositions soient présentés dans le même contexte qui comporte également d'importantes propositions de simplification administrative en direction des mineurs non accompagnés, lesquels continuent de se trouver dans un angle mort de nos politiques publiques ainsi avec Josiane Costes mon groupe espère ouvrir des travaux sur l'adaptation de la protection de l'enfance à ces nouveaux paradigmes juridique et sociétaux afin de renforcer l'égalité des chances, de tous les mineurs présents sur le sol de la République, nous sommes tout à fait favorable d'une part à ce que ce que le débat puisse se poursuivent dans un époux esprit de co-construction respectueux du travail parlementaire et, d'autre part à ce que tous les acteurs concernés puissent être associés à cette démarche, comme le permet la navette parlementaire sa lenteur a parfois des vertus, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Madame Corinne Imbert et vous avez 5 minutes. Merci madame la présidente, madame la présidente, monsieur le Ministre, madame, monsieur, les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons donc ce matin, la proposition de loi à l'initiative de notre collègue Josiane Costes les débats autour de la protection de l'enfance font souvent suite à des faits divers qui marquent profondément l'opinion publique, souvent sous le coup de l'émotion et sans véritable recul, c'est pourquoi je veux saluer le travail apaisée et délicat, réalisé par notre collègue auteur de ces propositions de loi nous donnant l'occasion ce matin de parler sereinement de ce sujet sensible mais passionnant, celle-ci à bord de 3 grands sujets : le 1er vise à renforcer la prise en compte de l'intérêt des mineurs, délaissée des pupilles de l'État. Cela se traduit par 2 idées fortes, à savoir renforcer la déclaration judiciaire de délassement et favoriser le recours à l'adoption simple en octobre dernier à la suite de la mission confiée par le 1er ministre nous vous avons remis monsieur le ministre, avec ma collègue députée Monique Limon, un rapport sur l'adoption, partant du constat que le nombre d'enfants confiés au titre de la protection de l'enfance étaient en augmentation et que dans le même temps, le nombre d'adoptions des pupilles de l'État était en diminution, c'est l'occasion pour moi de vous remercier à nouveau de la confiance que vous nous avez accordés à cette occasion, le renforcement de la procédure de déclaration judiciaire de délaissement était une de des préconisations de notre rapport, pendant longtemps il a été considéré que le maintien des Liens biologiques devait être la priorité toutefois depuis plusieurs années les considérer que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit prévaloir aussi l'épanouissement d'un enfant ne passe pas nécessairement par le maintien lien continue avec ses parents biologiques, les différents services de la protection de l'enfance en font quotidiennement le terrible constat et c'est l'occasion pour moi à ce moment de les remercier de tout le travail qu'ils ont fait et de du travail fait des dans les établissements et par les assistants familiaux à l'occasion de la pandémie que nous connaissons, partant du constat précédemment, la loi du 14 mars 2016 a instauré la mise en place de commissions d'évaluation de la situation du statut des enfants confiés les fameuses c'est 4 ans plus tard, un peu moins de la moitié des départements n'a pas encore procédé à la mise en place de cette commission, non pas par mauvaise volonté et parce que les services de la protection de l'enfance sont en tension, confronté à une augmentation du nombre d'enfants placés et à la diminution du nombre d'assistants familiaux recherchant sans cesse des places pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les enfants qui leur sont confiées et pour éviter justement des prises en charge dans les hôtels se pose en arrière-plan, bien évidemment, la question primordiale des moyens financiers dont peuvent disposer les départements pour assurer leur mission, un changement de statut pour un enfant, devenant à leurs pupilles et adoptable adoption simple apparaît évidemment comme une possibilité sécurisante à la fois pour l'enfant et pour les parents, historiquement, vous le savez l'adoption simple a vu le jour : plus d'un siècle et demi avant l'adoption plénière, mais nous savons que la très grande majorité des candidats à l'adoption, souhaite une adoption plénière, alors que le profit des enfants placés et des enfants, a adopté a profondément évolué ces dernières années, ainsi la proportion d'enfants dits à besoins spécifiques en raison de l'orage de leur profil psychologique ou de leur handicap, a fortement augmenté, rendant il faut bien le dire, leur adoption plus délicate, pas sans conséquences pour les services des conseils départementaux qui sont les acteurs incontournables de la protection de l'enfance, la pédagogie et l'accompagnement des candidats à l'aube, options sont des vrais enjeux, vous l'avez rappelé monsieur le Ministre. dans le même esprit, il serait pertinent de favoriser et de formaliser le parrainage afin de répondre à la diversité des profils d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, le 2ème sujet que cette proposition de loi abordé la prise en charge des mineurs au-delà de leur majorité les conseils départementaux ne sont pas insensibles évidemment à à ce sujet, à cette question, ils accompagnent régulièrement des jeunes majeurs, notamment quand ils sont en cours d'études, quand ils sont en apprentissage à l'inverse, il faut bien le dire, et notre collègue rapporteur de la commission des affaires sociales, l'a rappelé il y a des jeunes qui souhaitent évoluer de leurs proches et va évoluer, pardon de leurs propres ailes dès leur majorité et ne veulent surtout plus être accompagnés par les services de la protection de l'enfance, il nous faut peut-être accepter la diversité des situations, enfin le 3ème sujet de cette proposition de loi concerne les mineurs isolés étrangers, la plupart des départements ont été confrontés à une arrivée massive de mineurs non accompagnés, il est à noter quand même que depuis la mise en place du fichier bureau biométrique que nous attendions et que nous souhaitions au Sénat cette ce nombre d'arriver, a été a stagné, du moins sans diminuer, il a au moins, ils l'ont installé en Charente-Maritime, afin de faciliter la démarche administrative et les démarches administratives, au moment de la majorité pour ces mineurs non accompagnés et de l'arrêt de la prise en charge par le conseil départemental, nous avons fait le choix de travailler étroitement avec les services de l'État pour anticiper leur sortie du dispositif dans les meilleures conditions et d'éviter toute sortie sèche, nous l'avons vu cette proposition de loi balai plusieurs champs de la protection de l'enfance et je partage les propositions favorisant l'adoption simple et le parrainage : je préfère attendre et revoir ses sujets à l'occasion d'un grand texte sur l'adoption, rappelant, comme vous l'avez fait monsieur le ministre, que l'adoption, c'est d'abord donner une famille, un enfant, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur Jean-Yves Le pour 5 minutes. Merci madame la la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, d'abord, merci madame Josiane Costes pour cette occasion de d'échanger sur un un, un sujet majeur et sur plusieurs de ces aspects, en particulier sur le l'aspect que j'ai suivi plusieurs falloir des lois immigration sur les mineurs étrangers isolés, on le on le fait à un moment très très très particulier où la période de confinement à à à nous a malheureusement conduit à constater une hausse très importante des violences intrafamiliales et en particulier sur sur les enfants, si l'on regarde les les statistiques et communiquer ces ces derniers jours il est probable qu'énormément de familles seront déstabilisés par la situation sociale, leur situation d'emploi de revenus mais aussi la question de la capacité d'envoyer les enfants à l'école et et de faire face à tous ces défis qui rendront un certain nombre de familles déstabiliser avec des des capacités de, de, de, de, de violence et déstabilisation dans les familles important. La proposition de loi, tels que l'Inde et discutons aujourd'hui appellerait quand même quelques quelques remarques importantes car éloigné, hein, un enfant de de ses parents biologiques peut être parfois une nécessité, en particulier en cas de violence avérée, mais il faut faire en sorte que ce soit quand même le plus exceptionnel possible et en tant que possible, aussi réversible, parce que il ne faut jamais accélérer ce processus de destruction de famille et notre position est que le maintien du lien. Autant que possible et dans l'intérêt de l'enfant, c'est pour ça que l'actuel délai de délaissement de 12 mois nous semble un équilibre qu'il faudrait probablement pas remettre en cause 6 mois serait pour les enfants de moins de 3 ans, probablement avec un facteur de de de vecteurs de de graves dérives, quand on regarde ce qui peut se passer dans dans d'autres pays, il faut de toute façon, aider les parents qui sont déstabilisés dans un moment passager, ça peut arriver à aider à reconstruire les Liens avec leurs enfants, l'article 9 de la Convention des droits de l'enfant, ratifiée par la France en 1990 précise d'ailleurs que sauf malgré sont avérés, les États doivent veiller à ce que les enfants ne doivent pas être ne soient pas séparés de leurs enfants contre contre il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'aider les parents à garder autant que possible un lien avec leurs enfants, être même lorsqu'ils traverse une dépression, une maladie, un moment d'égarement même particulièrement grave et il ne faut pas que les conséquences soient systématiquement irréversible, c'est aussi pour la la raison pour laquelle nous nous nous opposerons à l'idée de la présomption de désintérêt pour les parents des mineurs étrangers isolés parce que c'est pas nécessairement une démarche d'abandon, c'est parfois dans un démarche de déchirement, la volonté de voir leur enfant échapper à une vie infernale la misère à l'exploitation, faudrait-il en plus qu'il y a une après une appréciation de cet acte qui engendre des conséquences sur la relation entre les parents et et leur enfant sur la question de la nationalité, quelques remarques. Quand je constate la manière avec laquelle on peut transmettre la nationalité française pour une adoption plénière. Totalement à l'étranger par rapport à l'adoption simple. Que vous proposez, je crois qu'il y a un petit décalage qui qui méritaient d'être travaillées, enfin il y a aussi une question de de 6 pour la la la nationalité française, une difficulté par rapport à la situation des, des, qui n'accepte pas une double nationalité, l'aide sociale à l'enfance est une mission essentielle et l'engagement de ces acteurs mérite d'être salué les statistiques qui tombent été donné tout à l'heure ne signe pas l'échec de la mais la difficulté de sa mission, et en particulier pour les jeunes étrangers, la question de la rupture après 18 ans, quelle différence entre un. Jour de plus, c'est un jour de moins la raison pour laquelle on fait les tests osseux aucun, nous avons tous été parents ici et nous savons que, du jour au lendemain, ben, les jeunes, ils ont aussi besoin d'accompagnement. Et c'est encore plus vrai pour ceux qui ont eu une enfance particulièrement compliqué, c'est la raison pour laquelle l'une des difficultés aujourd'hui, c'est cet accompagnement après 18 ans, est ce que vous proposez nous semble aller dans, dans, dans le bon sens parce que vous essayez d'y répondre, simplifier les parcours administratif, les questions d'éthique de séjour est essentiel, rejeté les tests se aussi regretté, je dois regretter à ce moment-là, à cette période du débat que d'opposition dans cette enceinte sur les mineurs isolés étrangers au moment de la loi asile immigration n'aient pas été bons, parce que nous avons fait une coupure à 18 ans qui qui nous permet, pas ensuite de donner un maximum de sens à ces jeunes qui ont pourtant été aidé avant 18 ans, enfin la zone doit être resté une politique nationale une priorité nationale, ça a été dit et elle a besoin de moyens en particulier pour accompagner les familles, les familles d'accueil, en tout cas merci Madame Coste pour cette cette démarche En plus, sur les 10 secondes qui me laisse Madame Monsieur le Ministre, je voudrais vous vous interrogez sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce qui est débattue dans la PPL mais qui me semble important, je ne veux pas évoqué directement le débat de la GPA mais les restrictions de circulation en Europe, dont les conséquences dramatiques pour les nouveau-nés le départ GP en particulier en Ukraine qui sont privés de l'accompagnement de leurs parents au moment où ils ouvrent les yeux sur le monde, faut-il Monsieur le ministre, pour des raisons morales d'éventuels qui un un éventuel appel d'air priver ses enfants de la chance de pouvoir être accompagnés de leurs familles au moment où ils ouvrent les yeux sur le monde, ça n'a rien à voir avec le débat d'aujourd'hui, mais c'est une question quand même préoccupante pour un certain nombre d'enfants français qui qui sont seuls à l'étranger aujourd'hui. Merci. La parole est maintenant à monsieur Guillaume Chevrollier vous avez 5 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme un certain nombre d'orateurs je voudrais commencer par remercier l'auteur de cette proposition de loi notre collègue Josiane Costes qui pose les différents enjeux, de la protection de l'enfance de façon éclairée, il me semble très positif et encourageant de discuter aujourd'hui ensemble au Sénat d'un sujet aussi vaste que difficile entre la la sortie de l'aide sociale à l'enfance où la situation, les mineurs non accompagnés d'autant qu'il est terriblement d'actualité puisque le confinement lié au coronavirus a constitué pour certains enfants à risque de maltraitance et a mis en lumière les difficultés des violences intrafamiliales la raison d'être de cette proposition, et donc de promouvoir un recours plus précoce à l'adoption simple d'enfants mineurs dont les parents sont défaillants, mais toujours vivant en pratique la loi rend l'adoption des enfants pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance très difficile, ce qui les expose à évoluer dans les structures peu propice à la mise en place de projets de vie stable et structurant ou de projets éducatifs afin de remédier aux complexité procédurale actuelle et de proposer une alternative davantage pérennes, le texte entend faciliter l'adoption de ces enfants mineurs ont la forme simple. C'est géré notamment de d'accélérer la procédure de déclaration judiciaire le délaissement parental dans le but d'offrir le plus tôt possible une prise en charge pérenne des enfants via l'adoption, je suis de l'avis du rapporteur, la précipitation ne semblent pas adaptées à des enjeux aussi décisif d'autant plus dans le contexte particulier de flou autour de la procréation médicalement assistée et de l'adoption par les personnes de même sexe il est indiscutable que notre rôle est de protéger les enfants et je suis que conscient que certaines situations familiales sont dramatiques, mais l'enfant ayant quasiment toujours intérêt in fine et à maintenir des Liens harmonieux avec sa famille naturelle empêche une amélioration semble excessif et nuire à l'intérêt de l'enfant, selon bon nombre d'acteurs spécialisés dans la protection de l'enfance il faut préserver autant que possible ce lien parents-enfants : les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, plus tôt on les accompagne plus en plus on augmente leurs chances de remplir pleinement leur rôle éducatif et de prévenir l'apparition de de difficultés éducatives majeures : la ligne de crête de la protection de l'enfance, c'est de réussir à concilier l'intérêt de l'enfant le respect de ses droits et le respect des droits des parents. La lutte contre la pauvreté et, par ailleurs, un enjeu réel, je rappelle que 80 % des enfants en situation de placement viennent de familles vivant avec un revenu en dessous du seuil de pauvreté, cette lutte contre la pauvreté, fondamentale, notamment pour améliorer la prise en charge des mineurs placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, au-delà de leur majorité comme le propose le 2ème objet du texte dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement a élaboré un certain nombre de mesures pour éviter ces sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, elles sont en cours de déploiement sur le territoire et Valon, lui, à moyen terme, avant d'on allait bords et d'autres concernant la généralisation de l'accompagnement des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans, il est de la responsabilité des départements d'accompagner les jeunes de l'ASE arrivant à 18 ans, à travers notamment les contrats jeunes majeurs, or il ne s'en affranchissent pas tous de la même façon, de plus, ces contrats vont prioritairement à des jeunes qui ont un solide projet, or ce sont ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement, ce sont ceux qui n'ont pas de projet pour les acteurs du terrain, il ne faudrait pas soumettre l'accompagnement des jeunes au-delà de 18 ans un projet précis, mais à l'aboutissement de l'Éducation du jeune en tous les cas, il faudrait prévoir un accompagnement vers la sortie de la zone au moins un an avant sa majorité afin de construire avec lui un projet. Très rapidement, pour finir sur l'amélioration de la prise en charge des mineurs non accompagnés, il semblerait qu'il y ait une nécessité plus vaste de repenser le cadre d'accueil de ces mineurs non accompagnés qui est un sujet tout à fait important pour les conseils départementaux, malgré le fait, comme je l'indiquais que ce texte pose de bonnes questions, tout comme la commission, je voterai contre, étant donné qu'il n'apporte pas de réponse suffisamment globale et efficiente, je pense notamment que les familles ont un rôle à jouer, le confinement, j'en veux pour preuve l'école à la maison, que les parents étaient les premiers éducateurs des enfants et si les parents devenait le Centre des politiques éducatives, je suis convaincu qu'une réflexion doit être menée autour de l'accompagnement à la parentalité dans la politique familiale, si nous accompagnons les parents nous ils accompagneront mieux leurs enfants, je vous remercie. Merci la discussion générale est Close. La commission n'ayant pas élaboré de textes, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initial, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'un espace réservé au groupe RDSE, qui a souhaité l'inscription de 2 points à l'ordre du jour, nous devons suspendre l'examen au terme du délai de 4 heures soit à 13 simplement petit rappel : nous avons une discussion qui doit s'y suivre celle-ci. Article 1, la parole est à Madame Josiane Costes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues permettez-moi de vous présenter cet article afin qu'il ne soit pas mal interprété la loi de 2016 a, comme vous le savez, transformer de la déclaration judiciaire d'abandon en la remplaçant par celle du délaissement parental en supprimant les l'élément d'intentionnalité qui résulter de la rédaction antérieure. La modification que je vous propose, aujourd'hui, consiste à affiner cet instrument en fonction de l'âge de l'enfant concerné par le délaissement parental afin de permettre aux institutions de protection de l'enfance de réagir plus rapidement au moment où l'enfant est le plus vulnérable en dessous de 3 ans les études de neurosciences souligne à quel point cette période et structurante pour le développement affectif de l'enfant, l'absence de scolarisation est également susceptible de renforcer l'isolement affectif, lorsque les parents font défaut, il n'est rue donc nécessaire de réduire la période de délaissement susceptibles de déclencher cette procédure judiciaire, nous connaissons tous les bouleversements que peuvent induire une licence pour les parents, mais il ne s'agit pas ici de retirer de sa famille, un enfant parce que l'un de ses parents seraient Athènes d'une dépression passagère nous disposons en réalité déjà du recul de la jurisprudence civile appliquée à la déclaration d'abandon comme indicateur et cette jurisprudence apparaît particulièrement protectrice de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi, les juges ont parfois écarté une telle procédure lorsqu'elle aurait paradoxalement conduit à une loi ni l'enfant d'une famille d'accueil, à laquelle il était très attaché, lorsque tous les critères de l'abandon était retenu en outre la jurisprudence garantit également que mineure délaissée qui ont été pris en charge par un autre par un autre membre de sa famille par exemple, les grands-parents ne puisse faire l'objet de cette procédure, en définitive, cette proposition vise essentiellement pour les enfants, ne rentrant pas dans les catégories, je viens d'évoquer et se trouve en véritablement délaissé accéder plus rapidement aux juges en raison de leur très jeune âge afin de se voir offrir plus rapidement un projet de prise en charge plus structurant et potentiellement une adoption en forme simple je vous remercie. Merci, nous passons à l'amendement numéro 10 présenté par Monsieur Bonhomme. Merci, on a un président. Oui, mon amendement vise l'article 1er qui de la proposition qui prévoit que la déclaration judiciaire de délaissement peut-être prononcé pour les mineurs de moins de 3 ans après un délaissement de 6 mois. Cette mesure ça s'inspire du système existant en Grande-Bretagne étant à loyer le plus rapidement possible les enfants les plus jeunes, de leur famille biologique. Lorsque celle-ci, en tout cas, est considérée comme pouvant être dangereuse pour l'enfant, donc il me semble que la durée de actuellement fixée à un an, doit être maintenu en effet divisé cette durée de moitié pourrait donner lieu à des dérives, notamment s'agissant du nombre d'enfants pour faire l'objet d'une adoption si cette durée de 6 mois pour délaissement était adopté. On peut se demander comment seront traités alors à l'avenir les situations suivantes les parrains, malades ou traversait une crise qui ne peut pas, pour des raisons de santé se manifester auprès de son enfant durant 6 mois. Alors la commission des lois, estimé que le délit de non-prise en compte pour constater le délaissement parental était un délai raisonnable qui permet de prendre en compte les accidents de la vie auxquelles peuvent être confrontés certains parents et donc il n'y a pas lieu d'accélérer cette procédure, mais plutôt de mieux l'appliquer et notamment détecter plus tôt les situations de délaissement grâce à un examen régulier des situations des enfants ensuite, mais je l'ai dit dans mon propos liminaire, il faut savoir que le lien entre délaissement l'adoption n'est pas automatique, tous les enfants délaissés ne devienne pas pupilles de l'État et toutes les pupilles et tous les pupilles de l'État ne sont pas nécessairement adoptables donc les raisons de la non-l'IT ne sont pas toujours liés à l'âge de l'enfant, ce sont les raisons pour lesquelles la commission. N'a pas adopté l'article 1 elle a émis un avis favorable donc à l'amendement de suppression de notre collègue François Bonhomme. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre. Merci madame la bas, la présidente, ce sera un avis favorable et pour globalement les mêmes raisons que le que le que le rapporteur, la procédure déclaration judiciaire délaissement parental a été créée, ça a été rappelé pour substituer à l'ancienne déclaration judiciaire d'abandon par la loi de de 2016 les objectifs étaient notamment de faciliter le recours à la procédure délaissement parental et de fixer des critères objectifs délaissement qu'soit centré sur la personne de l'enfant, plus de 4 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, le bilan plutôt positif puisque le nombre de demandes faites a plus que doublé et que le les rejets sont rares 32 pour 689 demandes sur l'année 2018, l'article 1er prévoit une nouvelle évolution des textes pour permettre un délaissement soit constaté au bout de seulement 6 mois pour les enfants de moins de 3 ans, ce qui nous paraît la même façon peu disproportionnée probablement inadaptées aussi, car les jeunes parents ou une jeune mère isolée peuvent être fragilisées par la naissance, mais c'est tout le sens de la protection enfance aussi de se ressaisir et c'est notre rôle d'accompagner d'étayer les parents en difficulté et de leur apporter un soutien approprié, donc il n'est pas souhaitable pour l'enfant de le couper de ses parents après seulement 6 mois, si, si, un travail éducatif peut en réalité être effectué et ça doit être, c'est par ailleurs une des mes ambitions qui nous anime, notamment dans le volet prévention, ça a été évoqué tout à l'heure, je pense aux 1000 jours au programme sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, donc aucune adoption pourrait être travailler sereinement et dans l'intérêt de l'enfant, les droits de la famille d'origine n'ont pas été prises en compte les textes actuels sur la déclaration judiciaire de délaissement parental sont équilibrés et répondent aux objectifs fixés en mettant au coeur de ces procédures, l'intérêt de l'enfant afin, pour autant, de répondre à votre préoccupation madame la la sénatrice un compromis, je crois, a été élaborée que vous aurez l'occasion de défendre et que nous aurons le plaisir de soutenir. Merci monsieur Yachvili, vous avez la parole pour l'explication de vote. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi effectivement je suis pas favorable à ce délai de, de, de 6 mois et je pense que oui, enfin nous allons voter, donc du coup, l'amendement de suppression, notamment parce que si moi, ce n'est, malheureusement, dans les faits et dans la pratique peu réalisable, moi je comprends bien le l'intérêt de l'objectif qui est encore une fois, l'intérêt supérieur de l'enfant, mais où il y a aussi une question de pratique, il y a aussi une question de réalités sur le terrain et je pense qu'il serait peut peut-être plus intéressant de s'assurer que les commissions d'évaluation de la situation du statut de l'enfant confié soient réellement mis en place dans les départements, puisque, a priori, c'est quand même pas le cas dans tous les départements, alors que ça date depuis la loi de 2016 et je pense que là il y a un vrai sujet, plutôt que de rabaisser ce délai à 6 mois, je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 10 avec 2 favorable qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, après l'article 1er nous avons l'amendement cette rectifié Madame Coste. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement rejoint la préoccupation exprimée à l'article 1er visant à adapter un peu mieux les procédures de protection de l'enfant en fonction de son âge afin de la compagnie au mieux son développement, les services d'aide sociale à l'enfance et la mort tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, un rapport établi après une évaluation pluridisciplinaire qui fait l'objet d'un examen au niveau de chaque département par une commission d'examen spécifique, il est donc proposé d'éteindre cette évaluation régulière au-delà de 2 ans jusqu'à 3 ans acheter théorique de la scolarisation en classe maternelle, je vous remercie. La commission a approuvé l'initiative de Madame Coste d'inclure les enfants de 2 à 3 ans dans le suivi opérer tous les 6 mois par les services d'aide sociale à l'enfance, donc avis favorable. Merci, Monsieur le Ministre. Avis favorable de la même fin. qui est contre, il est adopté, article 2 nous avons l'amendement numéro 11 présenté par Monsieur Bonhomme. Merci la la présidente. L'article de la proposition tant à renforcer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement depuis 2016, je rappelle que le constat a été fait que l'obligation de proposer aux parents des délaissant des mesures appropriées contribue à protéger les parents et non pas l'intérêt de l'enfant dans le cas d'un mineur de moins de 3 ans, la prise de décision du juge serait accélérée par la limitation de l'instruction par le juge a un mois, cette durée passerait à 2 mois pour les mineurs de plus de 3 ans donc cet amendement tend à supprimer l'article 2 qui aurait pour conséquence de priver l'enfant de ses parents temporairement empêchées, en effet, n'importe quel parent peut-être confronté à un moment donné à des difficultés passagères de durée variable sans pour autant souhaiter abandonner leur enfant. Merci, monsieur le rapporteur. l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant, la commission des lois, s'est donc prononcée contre la suppression de l'obligation de proposer des mesures de soutien aux parents, délaissant quant à la durée d'examen des demandes en déclaration de délaissement imposée au tribunal judiciaire un délai de 2 mois voire 2 pour se prononcer, semble irréaliste et peu souhaitables, le tribunal doit pouvoir réunir des éléments d'information, l'avis du juge des enfants et organiser un débat contradictoire, il a un va de l'intérêt de l'enfant et des droits de la défense, donc avis favorable à l'amendement de suppression. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Merci madame la présidente, ce sera aussi un avis favorable à cet amendement de suppression de l'article que vous demandez dont vous demandez la suppression, pardon, Monsieur le Sénateur, prévoit en effet de supprimer ce devoir d'apporter des mesures de soutien au aux parents, or pour caractériser une absence d'implication des parents, il faut nécessairement avoir donné aux parents la possibilité de s'investir dans le travail éducatif en leur donnant les moyens parce que. C'est pas facile d'être parent, on vous apprend pas être parent. Et on nous apprend beaucoup de choses dans la vie, conduire à traverser la rue et ça ne met pas être parent, il y a des parents qui sont de vulnérabilité de toute nature pas que social. De toute nature qui peuvent rendent difficile, difficile, l'éducation et il est important que nous soyons à leurs côtés pour les aider, voilà donc si rien n'est proposé, il serait, nous semble-t-il particulièrement abusif de prononcer un délaissement parental et ce ne sera en tout cas en aucun cas conforme à l'intérêt de l'enfant voilà cet article 2 prévoit par ailleurs à des traitements de mois, voire d'un mois, qui là aussi nous semble contraire, d'une part, à l'expérience des juges auxquels il faut laisser aussi peu de marge de manoeuvre ou pour apprécier les situations et puis aux intérêts des, des,

Qui est contre, il est adopté, l'article est supprimé, nous passons à l'article 3 avec l'amendement 12 présenté par Monsieur Bonhomme. Merci dans le président, c'est également un amendement de suppression de l'article 3 de la proposition promeut l'adoption simple auprès des parents souhaitant placer leur enfant auprès de la en vue d'une adoption, l'objectif serait de réduire le risque d'instabilité pour l'enfant pouvant résulter d'une reprise, il s'agit de laisser une place à la famille biologique, cet amendement supprime donc ce dispositif, ce sont les parents adoptifs qui doivent décider du type d'adoption qui choisissent pour leur enfant l'adoption plénière est la forme la plus protectrice d'adoption pour le nouveau lien familial, l'article 3 de la proposition de loi semble donc vouloir tenir compte voir imposer la décision des parents biologiques, la persistance du lien biologique peut avoir de graves conséquences pour l'enfant, notamment une incompréhension de sa situation entre la famille biologique et sa famille adoptive cette situation de perturbations chez l'enfant et constaté avec des familles d'accueil, en général, dans cette hypothèse, le maintien du lien entre les parents biologiques, tout au long de la minorité mène à des situations d'échec et parfois de fortes perturbations pour l'enfant. Qui, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, ce qui ce qui n'est pas souhaitable et je rejoins Monsieur Bonhomme sur ce point, c'est que ce soit les parents biologiques et qui choisissent le mois d'de l'adoption pour pour leur enfant l'adoption doit se faire dans l'intérêt de l'enfant et, selon le mot de qui lui est le plus bénéfique, c'est in fine et le Haut conseil de famille au nom de cet intérêt supérieur de l'enfant qu'il revient de décider alors la nouvelle rédaction proposée par Madame Cosse semblé un compromis acceptable, à la Commission, car le méthane avant le consentement des parents et non plus leur choix, donc je demanderais à notre collègue François Bonneau mais s'il veut bien retirer son amendement au profit de celui que va présenter Josiane Costes, qu'elle a donc réécrit. Merci, Monsieur le Ministre, Qui laissent leur enfant peut. Participer utilement. à la construction réussie du projet d'adoption, mais évidemment, ça ne peut pas être leur choix exclusif qui guide et ça ne peut pas être systématique, mais ça peut contribuer. à un projet d'adoption réussie, voilà et donc c'est pour ça qu'il faut laisser la possibilité et je crois que c'est tout le sens de l'amendement qui sera déposée par Madame la sénatrice, donc oui plutôt à une demande de retrait ou défavorables pour l'Allemande non de suppression afin de permettre que puisse ceci accroché un amendement de la sénatrice costaud auquel je serai favorable Monsieur Bonhomme. Vous avez demandes de retrait. écoutez à c'est avec plaisir, je suis pas toujours comme sur le fond mais Madame Coste propose un dispositif qui, quand même, par un compromis satisfaisant, je demande je j'accepte avec plaisir le retrait. S'il ne passe pas, sont donc à l'amendement 8 rectifié bis présenté par Madame Coste. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tenter de lever les inquiétudes exprimées par notre collègue François Bonhomme et d'autres d'entre vous sur ce cet article, l'article 3 de notre proposition de loi vise en effet à instaurer une relation de confiance entre les parents biologiques et les services sociaux, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, chacun d'entre nous peut imaginer l'état émotionnel très difficile d'un parent, constatant son incapacité à exercer son autorité parentale est amené à envisager l'adoption de son enfant par une autre famille, nous pensons que la possibilité ouverte par l'adoption simple de permettre à l'enfant lorsqu'il le souhaitera, d'explorer ses origines après s'être développé dans un univers familial beaucoup plus structuré, peut inciter davantage de parents biologiques en situation très difficile de faire ce choix-là dans l'intérêt supérieur de leur enfant l'adoption simple n'efface pas les Liens biologiques et permet même de conserver le patronyme d'origine de l'enfant, le recueil de la forme d'adoption sous d'être d'adoption souhaitées par les parents biologiques n'aurait aucune forme contraignante pour le conseil de famille.

les procédures d'adoption et de et de rendent l'adoption simple instauré par la loi de 2016 davantage qu'on puisse davantage y avoir recours, mais que les choses soient bien claires, ce n'est qu'une expression formulée, c'est bien le conseil de famille en dernière hypothèse au nom du seul intérêt supérieur de l'enfant, qui prendra la décision, ça, ça ne change pas et c'est cardinal et c'est important. Merci donc je vais mettre aux voix l'article 8 rectifié bis avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre l'article 3 est ainsi rédigé de façon à l'article IV avec une demande de parole de Madame Esther Benbassa. Merci madame la présidente, l'article 4 dans sa rédaction actuelle vise à encadrer les conditions de reprise par ses parents de l'enfant placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des formalités sont exigés, un entretien avec le tuteur de l'enfant et la convocation du conseil de famille nous pouvons hélas craindre qu'un telle dispositifs ne soient contre productive et stigmatise des parents ayant délaissé leur enfant alors que toutes les familles ayant eu recours à une telle procédure ne possède pas le même profil, tous les parents, délaissant endiguée mais ne sont pas forcément maltraitant, certains préfèrent confier leurs enfants à l'ASE en raison de problèmes sociaux, financiers ou encore sanitaires, or la maladie ou les problèmes d'argent peuvent parfaitement être passager, il ne serait donc pas compréhensible de refuser un retour simple des enfants au sein d'un foyer ayant retrouvé une situation dite normale, le droit positif et par ailleurs suffisamment protecteur dans la mesure où un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social des parents et de l'enfant et proposé pendant les 3 années qui suivent la procédure de délaissement, bien que nous partagions tous et toute l'objectif défendu par Madame Cosse, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne nous sommes pas que cet article soit de nature à en garantir l'effectivité merci. Merci madame je n'à Josiane Costes, vous avez la parole. Si madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le même esprit que les précédents ça cet article vise à mieux articuler l'intérêt supérieur de la vie de l'enfant et le droit de mener une vie familiale normale de ses parents, en renforçant les conditions de reprise de l'enfant par ses parents biologiques à l'issue du placement auprès des services de l'ASE, en effet, lors d'un placement auprès des services de l'ASE, l'enfant n'a pas la capacité de choisir et d'être maître de son sort, contrairement à son parent ça vulnérable vulnérabilité plus grande et de ce fait son intérêt supérieur nous paraît primer sur le droit à mener une fille familiale normale du parent la décision QPC à laquelle il est fait référence dans le rapport concernés en l'espèce un père biologique qui ignorait la date et le lieu de naissance de l'enfant et n'avait donc pas pu s'opposer au placement de l'enfant né sous X au service de l'ASE, il s'agit d'un cas de figure très précis, non représentative des situations donnant lieu au placement d'enfants auprès des services de l'ASE et l'équilibre trouvé par le Conseil constitutionnel face à ce cas d'espèce,

nous devrions aussi avoir une quasi-obligation d'avoir un avocat une assistance juridique juridique à la fois pour pour les parents dans cette procédure, mais aussi pour les enfants puisqu'on parle de la ville leur vulnérabilité des enfants, mais parfois les intérêts de l'enfant sont contradictoires, des intérêts de sa sa famille biologique et je pense que avoir une assistance juridique, un avocat obligatoire quasi d'office par pour pour ces ces procédures permettrait effectivement de régler un certain nombre de sujets, j'entends bien les arguments qui me disent que c'est l'ASE qui fait Office de protection de de l'enfant et qui mais je pense que, au-delà de ça, il faut que qu'il y a une assistance juridique importante et l'avocat peut permettre de faire cela, je vous remercie. Merci, nous passons à l'amendement numéro 13 présenté par Monsieur Bonhomme. Merci la présidente l'article 4 de la proposition renforce les conditions de reprise d'un d'un enfant placé un naze. à l'initiative de l'homme ou des 2 parents le droit positif prévoit que cette reprise peut intervenir sans aucune formalité, le renforcement de ses conditions de reprise serait justifiée par une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant, le dispositif proposé par cet article n'est pas à l'auteur des enjeux cet amendement tend donc à le supprimer à supprimer cet article en effet les conditions de reprise de l'enfance déjà strict et il serait souhaitable que l'accompagnement de du parent et de l'enfant, prévue à l'article L 224 précise du code de l'action sociale et des familles relève du juge des enfants et non pas du président du conseil départemental, en effet, la pratique

cet accompagnement devrait donc être une décision juridictionnelle connaissance prise du rapport de l'ASE et des autres intervenants qui assiste l'enfant y compris son avocat. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission. Alors l'article 4 vise à rendre plus difficile la reprise de l'enfant, remis à la The par ses parents en imposant de formalités, un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille dont on ignore d'ailleurs le rôle pourrait-il s'opposer au retour de la fin, je sais par an, ce dispositif est susceptible de rompre l'équilibre établi par l'article L 222 4 6 du code de l'action sociale et des familles, relevée par le Conseil constitutionnel, entre les droits des parents de dessin, c'est l'objectif de favoriser l'adoption, le délai de réflexion de 2 mois semble déjà bref au regard des conséquences de la décision prise de remettre son enfant à l'ASE donc avis favorable de la commission à l'amendement de suppression. Oui, la même façon et parce que c'était effectivement très convaincant, la peur du rapporteur et pour les mêmes raisons, ça sera un avis favorable à la suppression, effectivement, ça a été très bien rappelé depuis la loi de 2016 en cas de restitution d'un d'un enfant à ses parents, le Conseil des partants, le propose un appart, un accompagnement social, psychologique, éducatif. Du parent et de l'enfant pendant les 3 ans qui suivent la restitution de l'enfance, un dispositif qui nous semble approprié qu'il serait dommage de remettre en cause, voilà donc ce sera un avis favorable. Merci, je mets donc aux voix l'amendement numéro 13 avec 2 avis favorable qui est pour, Merci, je souhaitais au sujet de cet article, rappeler que la commission des affaires sociales, ne l'avait pas adoptés aux raisons qui l'était déjà satisfait en effet le droit en vigueur ne prévoit aucun nombre minimal concernant le les agréments l'assistant familial peut être agréés pour l'accueil d'un seul enfant. Merci, je mets donc aux voix, l'article 5 qui est pour. Alors, je vois des des mains qui se lèvent timidement je me voir l'article 5 après la prise de parole que vous venez d'entente de Madame la rapporteure donc. Pardon. Oui, monsieur le ministre. j'ai commencé le le vote donc normalement, vous ne pouvez pas vous exprimer mais donc je mise aux voix, l'article 5 qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté à l'article 6 nous avons une demande de parole de monsieur Xavier il madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai j'ai pas revenir sur l'ensemble de la discussion générale, où j'ai déjà pas mal parlé sur la compte la question des contrats jeunes majeurs, j'ai rappelé les chiffres, 70 % des jeunes sortent sans diplôme 40 % des sans domicile fixe de moins de 25 ans sont ont eu un parcours à l'ASE, monsieur le Ministre vous disait tout à l'heure 66 % des enfants sous protection de l'enfance ont déjà un an de retard à partir de la 6ème, donc conscients de cette réalité, le gouvernement a décidé de mettre fin à toutes les sorties sèches pendant la durée du confinement j'espère d'ailleurs pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, mais afin de protéger donc justement ces jeunes majeurs face aux risques auxquels ils sont exposés, vous avez rappelé monsieur le Ministre votre engagement afin d'éviter que les jeunes pris en charge par l'ASE se retrouvent à 18 ans, livrés à eux-mêmes sans ressources, sans logement, sans accompagnement, j'espère que vous nous donnerez peut-être des chiffres encourageants sur la contractualisation qui est qui est prévu avec avec les départements et les premiers résultats en tout cas de de de protection de de ses enfants, cette priorité est au coeur de la stratégie nationale de prévention que vous avez mis en place, de lutte contre la pauvreté et je m'en réjouis, le contrat jeune majeur fait dans un certain nombre de départements office de variable d'ajustement, la ministre Rossignol le disait en 2016, mais c'est l'angle mort des politiques sociales, la protection de l'enfance, et particulièrement la question des contrats jeunes majeurs, moi j'ai entendu en commission, que des enfants de 18. Temps avait envie de quitter très vite les institutions très vite l'ASE mais la question n'est pas une obligation, jusqu'à 21 ans, mais la possibilité pour les enfants qui ont besoin de pouvoir être suivie jusqu'à 21 ans, et encore une fois, à 21 ans, c'est pas la panacée, chers collègues, 21 ans, ce n'est même pas là, enfin on nos propres enfants, on les laisse pas partir à 21 ans de de chez nous, donc il y a une vraie réalité sociale de en tout cas tous ceux qui sont encore en études ne partent pas à 21 ans, et donc ils ont encore besoin d'accompagnement et besoin encore. De de de l'ASE, donc moi je, je suis bien sûr favorable à cet article que j'avais déjà pris cet article dans la PPL que que j'avais déposé en en juillet dernier, donc je ne vais pas me dédire sur sur cette. Cette proposition, nous ne pouvons plus accepter que des jeunes qui soient pris en charge par la les tout c'est enfonce qui soient plus fragiles dont le parcours fut si souvent difficiles soient jetés à la rue, à 18 ans, moi je suis dans un département qui a la chance de ne pas avoir de problèmes d'argent Les Hauts-de-Seine

Madame Josiane Costes, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame la présidente, moi je voulais insister reprend les propos de mon collègue Yachvili parce que effectivement ces contrats jeunes majeurs sont vraiment nécessaires, on n'empêchera pas les jeunes qui ont envie de partir de l'à 18 ans partir bien entendu c'est pas là le sujet, mais de nombreux jeunes ont besoin d'un accompagnement complémentaire, les chiffres ont été donnés en c'est aussi dans les EPM que j'ai eu l'occasion de visiter

c'est beaucoup trop jeune, même nos enfants qui vivent dans des familles structuré et et aimante et bien encadré à 18 ans, ils ne sont pas prêts à affronter la vie, donc des enfants qui ont subi subi parce qu'il s'agit de subir des parcours chaotique des parcours déstructurant, ils ont besoin de cet accompagnement alors justement l'adoption simple, ça serait un moyen de dégager des fonds puisque ça les conseils départementaux aurait moins d'argent à débourser et cet argent là, on pourrait le mettre pour l'accompagnement des jeunes après 18 ans, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Élisabeth Doineau. Oui merci, ce sujet me tient particulièrement à coeur, je pense que les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, en fait on les prive d'un choix et avoir le choix, c'est un luxe et ce luxe, il faut aussi leur offrir et la proposition qui est faite, c'est sûr, et est assez séduisante, mais je crois profondément que les jeunes qui ont été longtemps à l'aide sociale à l'enfance, ils ont envie parfois de perdre ce lien, je ne dis pas tout le temps, mais parfois de personnes, il faudrait leur permettre justement d'avoir ce choix de ne plus être en fait dans cette catégorie de jeunes et donc moi ce que je propose, c'est que justement, ceux qui veulent rester à l'aide sociale en France avec un contrat jeune majeur mais qu'il qu'il qu'il le reste mais pourquoi la barrière des 21 ans, vous l'avez dit, c'est parfois pas suffisant, moi je voudrais aussi qu'on voit le verre à moitié plein, on a des exemples plutôt que de dire : voilà, tous les mauvais exemples et là je viens de recevoir un Mail qui m'a dit qu'un jeune MNA va être donc soutenu par un contrat jeune majeur que que que évidemment je je vais favoriser dans mon département, il vient d'avoir le résultat de Parcoursup il va être admis en internat à Louis Legrand voilà des bons exemples, il faut les mettre en avant parce que nous avons dans nos départements de belles réussites des belles réussites et dans les études supérieures et aussi dans l'apprentissage et dans d'autres parcours et c'est par l'exemple qu'on arrivera à à à monter tout le monde vers le haut, et moi je pense qu'il faut aussi compter sur la réserve civique parce que du coup, on a vu pendant le Covid combien elle était précieuse cette réserve civique, il faut proposer à ces jeunes non plus d'être sous la responsabilité des départements mais sous la responsabilité d'autres institutions, d'autres organismes qui qui les accompagnerait et qui les porterait d'une autre façon que qu'avec des éducateurs, enfin je pense qu'on a vraiment les uns et les autres, sans doute, capacité essayer de travailler ce sujet est est pas là aujourd'hui, avec cette PPL mais je pense qu'il faut qu'on ait réfléchisse tous ensemble parce que ce qu'il faut donner à ces jeunes, c'est le choix et ce luxe du choix et ils ont le droit de l'avoir comme tous les autres enfants. Merci, la parole est à madame Michelle Gréaume. Mes chers collègues, pour moi, soutenir les jeunes de au-dessus des 18 ans, c'est très important, j'ai rencontré de nombreux jeunes qui arrivaient à 18 ans, malgré tout, il y a des familles, il faut savoir qu'il pouvait pu leur enfant. Il faut le savoir, des enfants sont pas forcément repris par les parents et il y a des jeunes qui arrivaient à 18 ans, ils veulent se battre pour sortir de la zone, sauf qu'ils ont besoin des aides, des aides techniques des aides financières, des aides pour le logement, il faut en être conscient, ne pas les laisser de sur le, sur le trottoir, c'est le cas de le dire parce qu'on a quand même beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui SDF qui sortent de la je rappelle et je vais faire un petit retour en arrière, je vais remonter très loin, j'ai remonté du temps où on a installé le RMI le RMI revenu minimum d'insertion, avant ça, les jeunes qui sortaient de l'armée ou qui sortaient de l'école avec un diplôme, avait déjà des ressources, on leur verser une une allocation chômage 2200 francs à l'époque, une fois que le RMI a été installée cette somme là n'a plus été donnée à ces jeunes à tous les jeunes Français que je parle, il y a eu aucune aide qui a été donné, on a tout intégré ça dans le RMI, puis dans le RSA, sauf que cette aide là aux jeunes également de rebondir là, moi je pense qu'il faut donner, il faut donner un espoir à ces jeunes de pouvoir pas avoir droit à une erreur, dites-moi, les jeunes de 18 ans, qui sont capables aujourd'hui de maîtriser leur avenir. Est ce que tous vos enfants à vous que vous avez eu vos petits-enfants, est ce que eux n'ont pas eu droit à une erreur, sauf que derrière il avaient avait des parents pour les aider, les soutenir alors moi je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir donner cette aide à ces jeunes et croyez moi c'est des jeunes demain qui ne tomberont pas dans la délinquance ou qui ne tomberont pas dans les mains de gens mafieux, tout ça parce que ils vont essayer de se battre plus que les autres à s'en sortir et pouvoir quitter le le l'aide sociale à l'enfance, alors soyons là pour les soutenir. Merci, Cet article, en fait, propose de rendre obligatoire l'accompagnement jusqu'à 21 ans, l'idée n'est pas de de dire que l'on arrête à 18 ans, de s'occuper des jeunes ou que l'on arrête à 21 ans l'idée et du caractère obligatoire et la commission des affaires sociales a préféré conserver le caractère enfin le le l'organisation sur une forme de souplesse, de dire que de de laisser les choses en l'état et de dire que, à partir de 18 ans les allées : accompagnement des jeunes qui, hein, le vol et je reprends les paroles de d'Élisabeth Doineau et de ce qui le nécessitent, peuvent être accompagnés par les départements sous la forme d'un contrat jeune majeur, donc elle s'est plutôt positionné sur le fait de ne pas rendre obligatoire cet accompagnement après 18 ans.

Qui implique le choix et je pense que la façon dont Xavier il y a, comme il y a à présenter notamment à présenter le sujet et la bonne, c'est-à-dire c'est c'est comment on accompagne ses enfants vers l'autonomie. Et donc cette question-là, elle se pose pas à 17 ans et 9 mois. Parfois, elle se pose sur le terrain 17 ans et 9 mois et ça aussi, il faut y travailler, mais en fait, elle se pose dès le début. Quand vous avez 66 % des gamins qui ont déjà un an de retard quand il rentre en 6ème. Là, déjà, on sent que ça. Porte atteinte à l'autonomie future quand 70 % des gamins ne vont pas ne font pas d'études supérieures, comprend bien, même si est une super, c'est pas l'Alpha et l'oméga il y a d'autres voies, mais on comprend bien que ça peut porter à la atteinte à leur autonomie, donc toute la question de l'accompagnement de ces jeunes vers l'autonomie, c'est tout au long du parcours travaillant sur l'éducatif sur l'accompagnement professionnel. Sur l'la intégration sociale plus large que ça se fait. Et permettez-moi madame la sénatrice moi aussi de remonter un peu en arrière : en 1989. Dans un autre Champ le handicap. Grand acteur Michel Creton. Fils polyhandicapé. Le pays n'avait pas à l'époque. pas beaucoup, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui la société change et c'est une bonne chose. D'instituts d'institutions. Pour les adultes handicapés.

Eh ben c'est pas résolu et en fait, vous avez des adultes qui sont dans des IME pour enfants. Beaucoup, qui donc excusez-moi les expressions que je suis un fervent partisan de la société inclusive mais occupent des places qui ne sont pas disponibles pour les enfants, et dont le handicap s'avère être plus élevé. Que les personnes de l'orage, qui ne sont pas nos institutions parce que évidemment l'accompagnement qui l'aurait fait n'est pas approprié. Donc moi je l'ai dit, je l'assume, ça m'a valu des inimitiés, mais je ne serai pas le ministre qui passerait l'amendement Creton de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, je pense que nous avons les moyens et que nous commençons déjà nous donner les moyens, je vais y revenir d'accompagner ses enfants vers l'autonomie, hé oui, nous avons une obligation de résultat, c'est insupportable d'imaginer qu'un enfant, qu'il soit passé par l'aide sociale en France ou pas, puissent terminer à la rue alors des avant ma nomination dès 2018 dans le cas de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, un volet spécifique a été dédiée à cette question-là. Avec l'attribution, je disais c'est des chiffes ces macro-ça a pas grand sens, mais de 12 millions d'euros qui ont été attribués au département pour pouvoir financer quelque chose de très important, le lien. Oui, il y a le logement, je vais y revenir, mais le lien maintenir un lien, vous l'avez très bien dit, enfin, à 18 ans, il y a pas de famille. Donc si tout d'un coup l'accompagnement social, les Liens qu'on a pu nouer avec son éducateur tombe. Mais c'est aussi des structurants. Que peut être l'absence de toi. Donc ça sert à financer ce maintien du lien notamment et alors j'ai des premiers chiffres qui nous ont été remontés par la délégation interministérielle de la prévention et de lutte contre la pauvreté, ce qui porte sur 67 départements parce que comme le rapporteur dans son propos liminaire l'évoquait, on a quand même un sujet de connaissance des données et qui fera partie de la réforme du gouvernement, ce que nous allons initier mais sur 67 départements l'année dernière, vous avez 14000 jeunes qui sont arrivés à la majorité, sur ces 14000 jeunes 10500 ont bénéficié dans le cas du plan pauvreté d'un accompagnement. Qui avait été élaboré d'ailleurs sur la base d'un référentiel qui avait été élaboré avec des jeunes, ancien. De l'aide sociale à l'enfance 10500 sur ces 10500 jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement à leur majorité, 7000 alors 5000 ça a été justement pour ce financement du lien qu'un éducateur puisse continuer à les suivre au delà de leur majorité 7000 ont eu un accompagnement financier pour trouver un logement. Alors vous allez me dire 7000 et 5000 ça fait plus que les 10500 que je vous ai donné mais c'est parce qu'on peut avoir une aide multiple

une fois leur majorité attente voilà mais donc voilà pour ses premiers ses 1er chiffre par ailleurs. Vous dire que redire que dans la la la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, mais aussi des choses en en place, je vous ai parlé tout à l'heure de l'expérimentation que nous faisons avec l'Union nationale pour l'habitat, des jeunes, l'usage. Où on a créé, on est en train de créer de façon explicite, un espèce de fond de ce la solvabilisation une espèce de subvention un peu coup de pouce comme ça pour les aider sur la partie logements

un accès prioritaire au logement étudiant le logement étudiant, ils le gardent pendant l'été parce que autrement, voilà, ils ont, ils ont nulle part où retourner, donc ils l'ont, pendant l'été, la bourse allait verser aussi pendant toute l'année. Et enfin, je l'évoquais tout à l'heure, la garantie jeunes doit être mobilisé, et puis, là aussi, il faut aller voir dans les territoires, moi j'ai été dans le Val-de-Marne. C'est notamment la vice-président de Santiago, que vous connaissez probablement. Mais, dans le Val-de-Marne. Quand le gamin à 17 ans, ils se mettent tous autour de la table. Alors il y a le département et puis les gens de Pôle emploi et puis il y a les gens de la préfecture et puis il y a les associations évidemment. Puis on commence à anticiper, et à se poser sur la situation des jeunes pour voir comment on va les accompagner vers vers l'autonomie, et c'est ça aussi, dont on doit s'inspirer pour pour améliorer et éviter les ruptures et améliorer la situation de ces jeunes, voilà

de façon très pragmatique, concrète, proche de la réalité de ses enfants, le fait de pouvoir tomber à la rue, plus que des mesures un peu couperet dont je pense une fois encore qu'il faut faire attention aux effets de bord voilà des effets de seuil. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur Philippe, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le Ministre, je vous ai en écouter attentivement dans votre explication et donc j'entends vos arguments, je voudrais simplement réagir rebondir à la fois à partir de l'exemple, vous avez pris à travers l'amendement Creton, sujet que je connais bien, dans le monde du handicap, mais d'une façon générale, sur la prise en charge sociale des situations particulières, des enfants s'arrêter notre problème ici et vous avez dans les mains une partie de la réponse avec votre gouvernement, c'est la l'administration la sur administration des systèmes qui fait qu'à un moment donné on fonctionne par case par situation par financement et on crée à travers ça, des ruptures de parcours de vie pour les différentes personnes concernées, que sur les personnes handicapées ou les enfants en difficulté un moment Creton, c'était une réponse adaptée à la situation du moment, mais aura été le vrai problème c'est la barrière des 18 ans, vous avez en main la possible de la faire sauter ces bailleurs de 18 ans, mais le problème c'est que, si elle existe, c'est pas comme ça, elle existe parce que, avant 18 ans, c'est l'état qui paye après 18 ans, ce sont les départements, et tant qu'on réglera pas cette simplification et cette souplesse administrative, on pourra voir les plus beaux discours, mais nous serons toujours là à rediscuter des mêmes situations en disons beaucoup de bonne volonté mais l'incapacité de faire parce que le vrai problème c'est la sur administration du système, c'est vrai pour le handicap et c'est vrai pour l'aide sociale à l'enfance. Merci. Bien, je vais donc mettre aux voix l'article 6 qui est pour. qui est contre,

Merci madame la présidente, j'ai essayé de me lever, vite, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous savons aujourd'hui que la départementalisation de l'aide sociale à l'enfance, produit des inégalités d'accès à l'adoption pour les familles en fonction de leur situation géographique sur notre territoire en l'absence d'une gestion nationale, cela participe à la déperdition démographique de certains départements et peut inciter des jeunes familles a déménagé pour tenter de satisfaire leur désir d'enfant par voie adoptive dans l'esprit de l'article 7 à suivre de la proposition de loi visant à renforcer l'égal accès à l'adoption des familles adoptantes, quelle que soit leur situation géographique sur le territoire, cet amendement vise à prévoir la mise en oeuvre d'une recommandation du rapport IGAS de 2019, contrôle des procédures d'adoption dans le département de Seine-Maritime de mars 2019, 2019 pardon et du rapport limon Imbert recommandation numéro 21 il s'agit en réalité de donner une base légale à la base nationale désagréments en vue de l'adoption, qui a été créé en 2013, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. permettant d'arriver à une meilleure mutualisation du dossier d'agrément entre départements qui permettrait aux conseils généraux départementaux aujourd'hui d'aller plus facilement rechercher des familles en dehors du département, lorsque cela est nécessaire, je pense en particulier aux enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire porteurs de pathologies ou de handicap ou encore un membre de fratrie. Ils représentent près de la moitié des pupilles de l'État mais correspondent rarement aux attentes des parents candidats à l'adoption, c'est donc plus difficile de leur trouver une famille : il s'agit d'un domaine sensible, celui des données personnelles et nous n'avons pas eu le temps d'expertiser cette mesure aussi la Commission préfère demander l'avis du gouvernement, à vous, Monsieur le Ministre. Alors à vous monsieur le Ministre, l'accompagnement des projets d'adoption de faciliter les échanges. Combien de nous avons tous eu des histoires, un de ses parents, qui sont venus nous voir dans nos dans nos circonscriptions dans nos dans nos locaux pour nous dire : mais moi j'ai un projet mais je ça fait des années que j'attends et alors j'ai déposé dans un autre département, On sent bien qu'il y a besoin d'avoir un peu un pilotage et la fluidité national et un pilotage national pour autant et on le sait, ce ne sera pas suffisant à régler toutes les situations, mais notamment pour les enfants à besoins spécifiques, ça peut permettre de de faire se rencontrer un désir et d'enfants et un, et un besoin de de parents, voilà donc ce sera favorable. Monsieur le rapporteur, vous suivez l'avis du gouvernement. Très bien, donc je voix l'amendement 9 rectifié avec 2 avis favorable qui est pour, qui est contre, il est adopté l'article 7 qui est pour,

Qui est contre, il n'est pas adopté, je mais ou l'article 10 qui est pour. Le même vote oui même vote, donc il n'est pas adopté, j'ai mis aux voix, l'article 9 et Madame, Esther Benbassa à la parole. Merci madame la présidente, le présent article 9 vise à limiter le montant de la part des allocations familiales versées à la famille en cas de placement de l'enfant auprès de l'eau, de l'aide sociale à l'enfance dans le droit positif lorsqu'un enfant et placer les allocations familiales sont en principe perçues par les services de l'ASE, la loi prévoit toutefois une dérogation à ce principe, lorsque l'enfant fait l'objet d'une me dit mesures judiciaire le juge peut alors décider de maintenir le versement de ces allocations à la famille, dans le cas où celles-ci participent à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de celui-ci dans son foyer. Dans ces cas spécifiques, la retenue partielle des allocations familiales ne saurait être justifiée appropriée au pertinente par ailleurs, nous ne saurions ignorer que nombre de familles des laissant et je mets délaissant dans la crise sanitaire liée au Covid 19 a davantage en avant cette dimension dans les foyers modestes en attestent les besoins croissants d'aide alimentaire dans les familles, au regard de la conjoncture actuelle, il semble qu'une telle disposition viendrait fragiliser encore plus les familles déjà paupérisé, il ne semble donc pas nécessaire de modifier la loi en vigueur, je vous en remercie. Merci Monsieur Bonhomme, vous avez la parole. Monsieur Bonhomme. Oui. Vous avez demandé la parole monsieur bonhomme non ah pardon, vous aviez levez la main, monsieur Yachvili, vous avez la parole. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors moi je suis un peu embêté parce qu'effectivement, dans ma proposition de loi, il y avait cet article, mot pour mot, et donc c'est difficile pour moi de dire que je ne vais pas voter cet article et pourtant, et pourtant j'ai évolué sur le sujet en un an et je pense effectivement que, il faut laisser le juge jugé et décidé de de cette suppression d'allocations familiales, puisque, encore une fois, on risque de précariser un peu plus les familles et de, de, de supprimer le le retour éventuel dans les familles et donc j'ai changé d'avis et donc je voterai contre cet amendement. cet article pardon. Merci, alors, nous passons à l'amendement numéro 4 avec Monsieur le la les, les, les, les interventions précédentes : il nous semble logique, c'est vrai, les choses sont déjà d'endroits, simplement nous il nous semble utile de laisser

dans son bien avec l'enfant, donc voilà c'est un amendement de de suppression. Merci, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission. C'est. Ah, c'est Madame Madame, la rapporteure. La commission des affaires sociales a émis des réserves sur cet article 9 qui propose que l'attribution des allocations familiales dues au titre de l'enfant placés ne puisse être maintenu à la famille, sur décision du juge qu'à titre partiel, il ressort des chiffres que nous avons obtenu qu'il n'est pas systématiquement déroger aux principes posés par la loi qui prévoit que les allocations familiales sont versées à l'ASE lorsque l'enfant est placé et que, par dérogation, elles peuvent être maintenus par le juge à la famille si celle-ci participent à la prise en charge de l'enfant ou pour favoriser son retour dans le foyer, il semble donc préférable de laisser le jus au juge le soin d'apprécier chaque cas les situations familiales et les raisons du placement pouvant être très différentes, en outre, je rappelle que l'allocation de rentrée scolaire n'est plus versée aux familles qui ont un enfant placé depuis la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, cette allocation est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant, date à laquelle le pécule lui est attribué. L'avis de la commission donc est favorable à la suppression de sa cet amendement qui demande la suppression de cet article, merci Monsieur le Ministre. La de la même façon, ce sera un avis favorable à la cet amendement de suppression. Plaine. Jugement l'appréciation de la situation au juge, pardon pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de famille pareil qu'il n'y a pas de situations pareilles. Que faisons-nous d'une d'une fratrie par exemple ou un enfant serait confiée, mais pas les autres et il y a déjà des difficultés sociales et alors quoi, on enfonce encore plus la famille. Et on empêche possible retour si tant est que ce soit dans son intérêt bien sûr de l'enfant dans sa famille non, voilà, il faut vraiment laisser l'appréciation au juge parce qu'une fois encore, il n'y a pas de situation pareille et il faut prendre en en compte la situation familiale, voilà donc favorables à cette suppression, merci, je mets donc. Aux l'amendement numéro 4 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre. Il est.

oui, nous sommes à l'amendement numéro 4 présenté par Monsieur le comte, qui est un amendement de suppression, donc qui est pour oui qui est contre, il était adopté, et l'article est supprimé. Il faut être très attentif merci article numéro 10 Madame Josiane Costes, vous avez la parole.

de contacts dématérialisé avec leur famille d'origine qui est souvent une réalité suffit à leur apporter la protection nécessaire qui convient à l'orage, l'amendement 21, précise le dispositif initial et vise à instaurer une présomption d'impossibilité d'exercer leur autorité parentale pour des parents située à l'étranger, cette disposition ne vise évidemment pas les jeunes gens étrangers venus en France pour des études correctement d'aussi domicilié et pris en charge par des membres ou des proches de leur famille, elle vise au contraire à mieux protéger les adolescents arrivés sur notre sol au terme de parcours dangereux fragilisée par cette expérience et par l'absence de protection et de prise en charge par un adulte digne de confiance, une fois arrivés sur le sol français, il s'agit simplement de prendre acte de leur isolement et de la VUB vulnérabilité qui en découlent. Quel est l'avis de la commission. l'objectif est ici toujours de faciliter la délégation au service de l'ASE de l'autorité parentale exercée sur les mineurs isolés présents sur le territoire, mais malgré la réécriture proposé c'est un avis défavorable car cette disposition présente toujours de sérieuses difficultés, l'avion, un Buzz en commission l'innovation proposée particulièrement attentatoire au droit des parents de ces enfants qui risquerait de se voir systématiquement retirer l'autorité parentale, on ne peut pas déduire du simple éloignement géographique, il y a des conséquences aussi définitives sur l'autorité parentale, d'ailleurs, les acteurs de terrain nous ont confirmé que certains parents de MNA connaissent voir souvent soutiennent le parcours migratoire de leur enfant, donc rédigé bien trop largement cette disposition s'appliquerait abusivement aux enfants de tous les Français de l'étranger qui réside dans un autre pays il s'appliquerait de même aux jeunes étrangers qui viennent d'être en France, Anne année de stage ou un échange scolaire reste préférable de s'en tenir au droit en vigueur, il faut laisser pleinement le juge apprécie au cas par cas, si l'éloignement rend ou non, les parents incapables d'exercer l'autorité parentale, sans créer de nouvelles présomption juridique, donc avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Avis défavorable pour les mêmes habits défavorable madame Michelle Gréaume, vous avez la parole. Merci tout à l'heure, j'ai entendu dans le rapport qu'on parlait de délaissement qui avait pas qu'il fallait faire attention justement au délaissement pour les enfants qu'ils arrivent en France, de l'équipe moins étrangers sauf que, il y a aussi les enfants qui sont arrivés en France qui sont enfants, on peut parler délaissement parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qu'on a obligé à prostituées en passant par pour la frontière, donc je pense que ça pourrait aller les protéger également

parce que bon, déjà j'ai exprimé tout à l'heure dans la discussion générale qu'on ne pouvait pas préjuger du fait que, parce que que que c'était un désintérêt d'avoir finalement envoyé ou faire en sorte que son enfant soit en France pour échapper à une situation particulièrement difficile dans le pays d'origine, donc considérer après que les parents se désintéresse et faciliter ça, ça nous semblait déjà un peu difficile mais alors avec la proposition qui est faite, maintenant on ajoute le risque c'est que on ne peut considérer que toute tout Français qui habitent à l'étranger et qui envoie son enfant en France va se retrouver dans cette situation, alors bon, on peut encore débattent du 1er thème alors le second, c'est quand même un risque en plus qui me semble pas raisonnable de, de, de, une disposition qui me semble pas raisonnable de prendre, dans, dans, dans,

se pencher sur les critères d'évaluation de l'isolement des DNA conduisant à leur protection et notamment, c'est l'un de 2 de ces critères, parce que cette évaluation est et bien trop souvent subjective conduit à des recours massif au TA et je pense que ça c'est aussi un des sujets sur lequel nous devrions débattre prochainement. Merci, je mets donc au. Oui, oui, merci, je vais mettre aux voix l'amendement 21 rectifié avec 2 avis défavorable, défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté, je mais ou l'article 10 qui est pour. Ce qui est contre. Il n'est pas adopté, je me voix l'article 11 qui est pour. Nous sommes à l'article 11 qui est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté mais je vois l'article 12 Madame Josiane Costes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question des mineurs isolés étrangers ne bouleverse pas seulement les rapports entre État et départements mais modifie également la charge contentieuse au sein des juridictions lors des visites de terrain, nous avons évoqué avec des juges, la possibilité de concentrer le suivi de ces mineurs par les juges des enfants. Comme cela l'a été dit, malgré la grande mobilisation d'associations très engagé auprès de ces mineurs manquent souvent d'adulte de référence, nous pensons qu'il serait dès lors souhaitable de limiter le nombre de figures d'autorité autour d'eux et de confier le suivi judiciaire de leur prise en charge au seul juge des enfants, nous entendons l'argument de cohérence et la nécessité de préserver des blocs de compétences néanmoins vu l'importance croissante du nombre de jeunes concernés, il nous semble indispensable d'adapter toutes nos institutions et en conséquence, y compris l'institution judiciaire. Merci. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Tout simplement pour expliquer pourquoi la commission est contre cet article, c'est simplement le le juge naturel et le juge des naturel de l'autorité parentale et soumise aux affaires familiales.

Qui est contre. Il n'est pas adopté, nous en sommes à l'article 13 et l'amendement 19 rectifié bis Madame Coste. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la membre de l'article 13 et l'amendement 19 revêtent une importance capitale, il s'agit de faciliter l'ouverture de compte en banque pour les mineurs isolés étrangers afin qu'il n'aient pas à porter sur eux, de l'argent liquide en marchant, en liquide, les allocations qui leur sont versées pour survivre, comme j'ai expliqué dès la commission cela les expose à une grande violence, voire les pousse à avoir recours à la violence pour se défendre et cette violence, produit de l'insécurité qui ne convient à personne,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 après avoir échangé avec des associations, il est apparu que la difficulté de se faire accompagner par par un représentant légal constitue le principal obstacle je proposé donc de prévoir qu'il puisse le faire seul dès qu'ils atteignent l'âge de travailler dans le cas de contrats d'apprentissage après nos échanges en commission, la rédaction a évolué, il s'agit d'un point essentiel selon moi quand ils veulent travailler ces jeunes, ils ont besoin d'avoir un compte ouvert quand il va le contrat d'apprentissage, il y en a beaucoup qui veulent s'insérer, ils ont besoin d'un compte ouvert en banque

Monsieur le Ministre, ce droit de ce droit au compte de façon effective parce que je pense que c'est ça le c'est ça le sujet, en réalité c'est c'est pas tant le la question du droit au compte que de l'effectivité de pouvoir en bénéficier effectivement et heureusement. Pas tout le temps de façon aussi dramatique que vous l'avez exposé effectivement la période de confinement, on a pu voir qu'un certain nombre de jeunes mineurs non accompagnés avaient des difficultés à pouvoir bénéficier des allocations diverses et variées dont il disposait alors pour autant, ça va être un avis défavorable à ce stade, dans la mesure où nous ressentons le besoin de travailler davantage sur le sujet ne je vous donne la position du du gouvernement, il nous sommes d'une part que cet amendement. Crée tout de même une discrimination entre mineurs étrangers mineurs français parce que ça sera les seuls mineurs étrangers qui pourront bénéficier de cette cette disposition oui qui sont confrontés effectivement et des difficultés que d'autres ne n'ont coup, je vous le concède aisément, mais la réalité du droit, hé bien celle-ci. Par ailleurs, en France, le régime de l'administration légale des biens par les titulaires de l'autorité parentale est un système de représentation et c'est là dessus probablement à travailler de notre côté, avec la Fédération française des banques, notamment la démarche accomplie par le représentant légal pour demander l'ouverture d'un compte au nom du mineur n'est pas un simple accompagnement c'est représentant légal, pardon, qui demande l'ouverture du compte et avant 16 ans c'est un le représentant légal qui le fait fonctionner avec une exception quand même qui sont les déposent sur un livret d'épargne va donc dans ce contexte nous paraît important de conserver une cohérence dans les règles qui régissent ce régime de protection des mineurs à fortiori des mineurs étrangers. ça ne nous sommes pas devoir être traité au sein de la procédure particulière du du droit au compte, mais une fois encore, nous partageons l'objectif donc ça sera un avis défavorable de la part du gouvernement, j'ai bien entendu la vie de la de la Commission nous engageons en tout état de cause, quelle que soit l'issue de ce vote à travailler pour aller vers une plus grande effectivité de de ce droit au compte, dans les faits, voilà. Merci monsieur Yachvili, vous avez la parole. je, je comprends effectivement les les problématiques et et la galère que aujourd'hui ces jeunes peuvent rencontrer pour accéder aux comptes dans la plupart des banques, on demande le titre de séjour, quand on est mineur non accompagné, on n'en a pas, il faudrait effectivement que le simple passeport puisse puisse se suffire mais on voit bien que, à la fois il y a des blocages des banques il y a une il y a aussi un refus systématique quasiment des banques pour pour ses comptes, donc c'est un vrai sujet, moi je ne voterai pas cet amendement parce que j'entends aussi la l'engagement du ministre, de travailler avec avec Bercy avec les banques pour pour essayer de trouver une solution pour régler cette situation donc je ne voterai pas mais je, je pense que c'est un vrai sujet et je remercie notre collègue cost d'avoir mis en lumière cette cette Monsieur le comte, vous avez la parole. Qui ont. Droit à une bourse Cruz qui, à cette période de l'année n'ont pas perçu un Euro de cette bourse par ceux qui n'ont pas pu ouvrir de compte bancaire parce qu'ils sont mineurs. C'est un sujet majeur sur lequel oui, on nous dit depuis des années, qu'il faut qu'on va travailler non vous votez maintenant et et je ne suis même pas sûr, monsieur le rapporteur, que ce soit juste une question d'effectivité puisque jusqu'à présent le droit juste refusé dans le cas des mineurs. Alors que faire si l'amendement de de Madame Costes, passe le mien tombe et l'amendement de la Corse, il est finalement moins dur puisqu'il a, en gros, il prête, il pose le postulat que le droit au compte est effectif, ce qui à mon sens bon est discutable, mais si passe, il faut aussi qu'il soit possible pour l'les l'les mineurs français qui font des études supérieures, donc je propose, monsieur le rapporteur, un sous-amendement à l'amendement de Madame Coste qui supprimerait et ça répondrait à l'une de vos observations, monsieur le Ministre, qui supprimerait tout simplement le mot étranger dans l'amendement de Madame Coste. Non, mais il s'agit d'une rédaction différente, donc je pense que le mien tombera automatiquement par quand je propose un sous- amendement pour supprimer le le le la l'adjectif étrangers à mineur dans dans cet amendement, de manière à gérer tous les cas. Monsieur le comte nous sommes dans la discussion de l'amendement, donc on ne sous-amende pas, à ce moment-là, c'est un petit peu tard Madame Coste. C'est un sujet absolument majeur, moi je vis dans un territoire où en étant où il y a des offres d'emploi disponibles ou on n'arrive pas à recruter dans l'hôtellerie, dans la restauration dans le bâtiment où on a des jeunes qui veulent s'impliquer qui veulent signer des contrats d'apprentissage et ils ne peuvent pas le faire, ils ont des problèmes pour se faire verser leur c'est c'est c'est dramatique alors les employeurs sont très mécontents dans mon département, parce que nous n'avons pas de chômage, nous avons des postes disponibles, au contraire, les jeunes qui veulent s'impliquer s'insérer dans la société que c'est donc moi ce que je proposerais, c'est peut-être réécrire voir si vous ne pouvez pas est ce que le gouvernement ne peut pas améliorer l'écriture de mon amendement pour que cet amendement puisse passer parce que c'est vraiment essentiel, c'est essentiel. Le président a demandé la parole, elle vous est donnée. qu'il n'était pas possible de déposer un sous-amendement lors de la discussion d'un amendement chez l'honneur de vous demander en vertu l'article du règlement, cela vous paraît justifiée, moi je considère que justement dans ce débat très riche, il est apparu qu'il y avait un intérêt à supprimer ce mot étranger parce que comme le dit mon collègue Leconte avec force, qu'est ce que vous voulez, des jeunes qui ont des bourses et qui ne peuvent pas les recevoir, c'est quand même absurde cette situation-là, je crois que, ici, tout le monde comprend. ce sujet donc voilà c'est un sous-amendement et moi je demande madame la présidente, que vous vouliez bien soumettre au vote ce sous-amendement avant l'amendement comme il est logique. Aurais bien volontiers, monsieur Sueur compte, je leur ai sous les yeux, ce qui ne devrait tarder. Oui,

Je vais demander au rapporteur son avis. Merci, monsieur le rapporteur. Voilà, nous avons un sous-amendement numéro 23 présenté par Monsieur le comte. Ce sous-amendement concerne je comprends le collègue sénateur des Français de l'étranger,

il me semble inutile à l'État bien sûr qu'il y a possibilité de sous-amender comme la mais je crois qu'il est inutile, puis, d'autre part je rajouterais qu'à ce niveau de la discussion législative, nous sommes dans une PPL et donc au début, on va voir si elle est, elle est intégrée à la suite des éléments positifs qui sortiront de cette PPL sont intégrées à un futur PJ du gouvernement ou compléter à l'Assemblée nationale, un petit peu plus mais en l'état actuel, il me semble qu'il ait un petit peu inutile. bien non, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, vous émettez un avis défavorable au sous-amendement de monsieur Leconte. Avis défavorable sous-amendement. Très bien monsieur le ministre.

Mais je m'engage de nouveau dans le cadre navette parlementaire ou de toutes les tous les projets qui ont été qui ont été lancées à travailler avec mon collègue au ministère de l'Économie et des Finances. Parce que vous avez bien compris qu'une partie de la réponse qui était aussi là-bas et et je j'en profiterai aussi pour appréhender, monsieur le sénateur, le sujet que vous avez bien voulu porter à notre connaissance, aujourd'hui, même si je suis assez d'accord avec le rapporteur, ils sont un petit peu, c'est un peu de sujets différents, me semble-t-il, mais je je vous, je vous assure, ici aussi

Qui est contre. Il n'est pas adopté c'est mais aux voix l'amendement 19 rectifié bis présenté par Madame Coste, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement

L'amendement est adopté et l'article est ainsi rédigé. Je vais mettre. On voit l'article non non non, d'abord, demandes de paroles de Madame Josiane Costes sur l'article 14. Si Si madame la présidente, monsieur le Ministre, mais mes chers collègues, je souhaiterais juste insister sur l'importance de cet article qui vise à garantir l'effectivité du droit prévu à l'article 27 de la Convention de 1951 relative aux réfugiés, tout en permettant une bonne administration, l'absence de titres d'identité reconnu comme authentique complexifie en effet toutes les procédures administratives et judiciaires dans les États de droit comme le nôtre, reposant sur des preuves écrites, il s'agit à la fois d'une perte de temps pour la personne concernée et pour l'administration, l'objectif de cet article était donc de permettre à toute personne se trouvant sur le territoire français d'être fixé définitivement sur l'authenticité attribués au titre d'identité dont elle se prévaut afin de limiter les recours inutiles les informations dont nous disposons nous laissent à penser que nos services diplomatiques et consulaires sont à même d'exercer ce contrôle rapidement et qu'une telle mesure ne comporterait pas le risque de rétention aux frontières ces vérifications ont déjà lié au moment de la soumission des demandes de VISA et ne concernerait donc pas les personnes en disposant, il s'agit également d'une proche d'une protection pour la personne titulaire de ce titre d'identité qui ne pourrait pas se le voir refuser par une autorité administrative non compétente, Merci. Nous passons à l'amendement numéro 16 présenté par Monsieur Bonhomme. L'article 14 de la proposition vise à permettre à la délivrance d'un certificat d'authentification de titres d'identité unique par les services de douane afin de simplifier des marchés illustratif des mineurs isolés étrangers, notamment en cas de dysfonctionnement de leurs services consulaires, cet amendement vise à supprimer cet article en raison du délai particulièrement long nécessaire à la délivrance de tels documents il résultera un risque de rétention accrus aux frontières. Merci, quel est l'avis de la commission. que le service des douanes des CIO délivrent des certificats d'authenticité, cela poserait plein de problèmes de difficulté d'abord la rédaction sur le de, de, de cet article est trop large, la portée juridique surtout et vraiment incertaine et ça poserait de cela poserait de très importantes difficultés opérationnelles, donc nous sommes favorables à la suppression de cet article. I : Monsieur le Ministre, pour les mêmes raisons, favorable à la suppression favorable très bien. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 16 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contraint, il est adopté, et l'article est supprimé, nous passons maintenant à l'article 15 avec une demande de parole de Madame Josiane Costes. Costes. Présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent article vise à faciliter l'accès des mineurs isolés étrangers au contrat d'apprentissage afin de leur permettre d'accéder plus rapidement à une autonomie financière et s'émanciper par le travail, dans beaucoup de départements comme le mien, je vous l'ai déjà dit des postes sont vacants dans de nombreux, nombreux secteurs il me parler dès lors qu'on aime convenable de refuser à des jeunes volontaires qui veulent s'intégrer, dit candidater au seul motif de leur nationalité, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub. qui à plusieurs reprises mon saisi depuis le début de mon mandat, sur des cas particuliers, par exemple, un collègue maire qui avait pris dans l'équipe des services techniques, un jeune homme qui a donné vraiment parfait de satisfaction et puis pour une histoire brumeuse de de documents d'identité s'est retrouvé avec en situation OQTF et puis la jeune femme qui souhaitait préparatrice en pharmacie qui allait tous les jours très régulièrement aux Restaurants du coeur, le jeune homme qui maintient l'équipe de foot locale et lui permet de faire de bonnes performances, bref rebondir sur tout ça et dire que, en effet, ces jeunes sont des forces vives pour nos territoires dans certains territoires ont grandement besoin dans le domaine professionnel mettant tous les domaines, en général, et que ce serait dommage, tous ces rendez-vous manqués, il faudrait plus de souplesse dans l'instruction de tous ces dossiers, voilà je voulais rebondir sur ce cas particulier, j'en profite pour présenter puisque j'ai la parole, mon amendement qui arrive en disant que j'ai demandé à ce que les possibilités de régularisation s'étendent, y compris aux jeunes qui sont aussi à en service civique voilà, bon, j'aurais pu, j'aurais aimé aller plus largement sur l'investissement associatif l'investissement sportif, etc en effet, nous avons parfois grand besoin de ces ressources que représentent tous ces jeunes, je vous remercie donc j'ai présenté mon amendement. Vous avez présenté votre amendement et nous allons avoir l'avis de monsieur le rapporteur. Alors nous comprenons ce que veut dire de notre collègue de sénatrice mais rendre pratiquement automatique le séjour, l'autorisation de séjour parce que on est inscrit au service civique vous avez compris les conséquences que cela pourrait avoir un amour. Pour ceux qui malheureusement font éventuellement de temps en temps, passer des heures, des des jeunes à une situation illégale au niveau du territoire, donc je crois qu'il faut laisser à mon avis, les préfets, agir sur le terrain, on comprend que, ici et là, il y a des cas, vous en avez eu, j'en ai eu aussi dans mon département, mais il s'agit de ne pas rendre automatique que cela parce que ce serait un petit peu le cas, il s'agirait pour les zones et les autres de savoir comme demandant à rentrer dans le service civique, on a forcément une autorisation de séjour et, malheureusement, nous aurions rapidement, beaucoup de jeunes qui rentreraient illégalement sur le territoire et je crois que, donc, pour cela, surtout pour cela, mais il y a aussi d'autres raisons, la commission est défavorable. Merci monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement. ça serait un avis défavorable sur le l'amendement et sur l'article aussi vous dire que. sur l'amendement la la suppression, effectivement, de cesser de ces 6 mois qui sont posées par l'article L 313 15 du ces aidants, ça permet d'encadrer la différence des types de séjours et sa suppression. En réalité, donnerait plus de latitude, je ne suis pas sûr que ce n'est pas les effets contre des effets contre-productifs par rapport à ce que vous cherchez, mais moi ce que j'aimerais vous dire c'est que. Dans le cas de la de la stratégie du gouvernement pour l'Asie et l'immigration, que vous évoquiez tout à l'heure monsieur le le sénateur, nous avons travaillé avec le ministre de l'Intérieur. Pour faire en sorte de mieux intégrer. Quand cela est possible, les mineurs non accompagnés qui sont sur notre sur notre sol. On s'est basé sur quoi je me suis basé en fait ce que j'ai sur ce que j'ai constaté dans les territoires parce que derrière les fantasmes que Brandt, un certain nombre Monsieur il y a des réalités humaines et territoriales. Et en fait quand on va sur le terrain, on voit des jeunes. Effectivement eu un parcours pour venir jusqu'à chez nous. Donc on la conscience la charge dramatique. On a des jeunes qui apprennent le français pour ceux qui ne sont pas francophone en quelques mois. J'ai envie de bosser, qui se mettent dans les filières d'apprentissage et dont Madame Coste, vous avez raison, un certain nombre d'entreprises sur les territoires n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir effectivement les embaucher. Je pense que la clé c'est l'anticipation. C'est comme pour ne ne jeune majeur de tout à l'heure. N'attendons pas le moment couperet pour commencer à se poser des questions et donc à laisser peser une épée de Damoclès sur la tête de ces jeunes moi je, on le voit dans leurs regards quand on va les voir. Et dans l'Oise, par exemple, sauf erreur, c'est toujours un doute, je me déplace beaucoup sur le terrain, donc je finis par un peu tout confondre même si chaque territoire est magnifique et spécifique mais, dans l'Oise, le préfet, le département ont passé une convention.

Mais on commence déjà évalue la situation, ça permet quand même de calmer un petit peu le les angoisses du jeune parce qu'ils voient une perspective et ça fait qu'à 18 ans, surtout on prend la décision et il y a pas 3 mois encore d'examen. Qui fait qu'on crée une rupture et que pendant les 3 mois, mais en fait, là aussi, on crée un trou et que la filière d'apprentissage par exemple, dans lequel il est doit s'arrêter parce qu'il y a plus de papier, etc, donc ça permet de fluidifier aussi les parcours et d'éviter de créer une rupture supplémentaire dans le cas du projet à l'immigration, vous reprendrez parce que que vous avez travaillé dessus monsieur le sénateur, semble-t-il, il y a une disposition qui prévoit que nous étendions par le biais d'une circulaire. C'est cela à l'ensemble des à l'ensemble du territoire ce type de procédure

Sont essentiels. Parce que, bien entendu, on peut toujours fait preuve de bonne volonté au cas par cas, on peut, par circulaire dire puisque des choses dérogatoire sont possibles aujourd'hui par du mauvais côté, dans ces cas-là, on le fait mais affirmer des droits. Parier sur l'intégration par le travail. C'est comme ça que la République s'est construit dans les moments où, à l'arrivée. Accueillir et intégrer. Cette proposition va dans ce sens-là, accompagné d'ailleurs par l'amendement, donc il me semble qu'il faut voter les 2. C'est vraiment un pari sur l'intégration républicaine. Sur le sens de la capacité, par le travail de s'intégrer. Et de le dire en disant c'est pas si vous êtes sages le préfet sera gentil non c'est d'affirmer de droit. Monsieur le comte madame sur le groupe, vous avez la parole. Merci monsieur le comte pour votre soutien, néanmoins, cet amendement a été essentiellement un amendement d'appel, je pense que vous l'aurez compris et c'est pour ça que je vais malgré tout le retirer mais Monsieur le mini, j'étais vraiment tellement sensible à ce que vous avez dit : je vous invite dans mon département, qui est la Nièvre parce que nous avons des cas concrets à vous présenter, nous aurions vraiment besoin de votre aide pour pouvoir les les résoudre ensemble, je vous remercie. Merci, il n'y a pas d'autres demandes de parole bien et je vais mettre aux voix l'article 15 qui est pour.

Qui est contre, Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, il y a-t-il des demandes d'explications de vote. Je n'en vois pas je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à apporter un cadre stable d'épanouissement et de développement aux mineurs vulnérables sur le territoire français, qui est pour.

Coste. La présidente, je voudrais remercier monsieur le ministre, je voudrais remercier, madame le rapporteur monsieur le rapporteur, et là l'ensemble des collègues pour la qualité des débats, merci. Merci le présent requis, a demandé la parole. mes chers collègues, vu l'heure qui suit bien avancé, les débats été fructueux, mais un peu long, donc je vous propose de remporter le second texte de l'espace réservé sur la proposition de résolution d'une assurance récolte au projet, un espace réservé du groupe RDSE, qui aura lieu le 24 juin dans les trouve un peu dommage de commencer avec il y a un texte de faire un peu léger et de revenir à mon après, bon, on a beaucoup de salles actuellement à faire, donc je propose donc qu'on maintienne de l'unité de l'analyse du texte et donc de remporter ce texte donc à la prochaine au prochain espace réservé du groupe. y a un président acte vous en ai donné l'examen de la proposition de résolution visant à encourager le développement de l'assurance récolte et donc retiré de notre ordre du jour. suivre suspende la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires, la séance est suspendue.